Monsieur le président, madame la Première ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, « La pire des choses serait de penser que nous, Européens, devrions être suivistes sur [le] sujet [de Taïwan] et nous adapter au rythme américain et à une surréaction chinoise Ces propos du Président de la République, à la suite de sa visite d'État en Chine, ont suscité un tollé international à la veille de manoeuvres chinoises sans précédent. Alors que les tensions sont maximales en ce qui concerne l'autonomie de l'île à l'égard de la Chine, nous regrettons ces propos maladroits, voire tout à fait dommageables, du chef de l'État. En affirmant que l'Europe doit incarner une troisième voie entre les États-Unis et la Chine, il a rendu notre positionnement diplomatique plus flou que jamais et illustré un « en même temps » qui, à l'évidence, n'est pas partagé par l'ensemble des pays européens, eux ayant fait le choix d'un partenariat américain en matière de protection ou de dissuasion. On peut s'interroger sur l'opportunité d'une telle déclaration à l'heure du conflit en Ukraine. En effet, nombreux sont les pays qui comptent sur la collaboration renforcée entre Bruxelles et Washington pour faire cesser cette guerre. Cette polyphonie ne peut que nous affaiblir Madame la Première ministre, ma question est donc double : la France va-t-elle lever toute ambiguïté sur sa position concernant Taïwan ? Et comment l'exécutif entend-il concrètement faire avancer l'idée d'autonomie européenne sans remettre en cause notre partenariat privilégié avec notre allié américain ?

C'est légitime, et il ne viendrait à personne l'idée de le contester. Le Président de la République l'a toujours dit : nous ne sommes pas à équidistance de Washington et de Pékin, nous partageons des valeurs. La relation avec Pékin s'inscrit dans un cadre européen très clair depuis 2019 : partenariat, concurrence économique et rivalité systémique. Nous voulons éviter une logique de confrontation bloc contre bloc. Taïwan, nous sommes opposés à toute modification unilatérale du, par la force. C'est une position claire et constante de la France. Dans le cadre de notre politique d'« une seule Chine », nous avons d'importantes coopérations avec Taïwan dans de nombreux domaines, et nous nous y tenons. Face aux défis qui se posent dans cette région, les Européens doivent aussi défendre leurs intérêts économiques de manière indépendante. Ils l'ont fait en développant des instruments de défense commerciale, précisément sur l'initiative de la France. C'est aussi le sens du, qui vise à diversifier nos sources d'approvisionnement. Au cours de son déplacement, le Président de la République a dit très clairement les choses au président Xi Jinping sur tous les sujets, dans le cadre d'un dialogue exigeant et franc, assez éloigné des polémiques. Eh bien,

J'entends que le Président de la République veuille faire de la souveraineté européenne une priorité. Erreur d'analyse ou faute tactique, peut-être ... Ses propos à son retour de Chine restent, pour autant, un magnifique cadeau diplomatique offert au président Xi Jinping.

Le ministre de l'intérieur, M. Darmanin, a menacé de manière à peine voilée la Ligue des droits de l'homme (LDH) de sanctions financières. Il a déclaré, pour être précis : « Je ne connais pas la subvention donnée par l'État, mais ça mérite d'être regardé dans le cadre des actions menées. » Madame la Première ministre, les choses sont claires, votre ministre de l'intérieur envisageait sans sourciller de remettre en cause les subventions à la LDH, car cette dernière avait exercé un rôle d'observateur et de vérification du respect des libertés et des droits à Sainte-Soline ou sur d'autres théâtres d'affrontements ou de tensions. Ces menaces sont d'une gravité insupportable. Pouvez-vous accepter qu'un ministre de la République envisage de porter atteinte à une association qui est l'honneur de cette dernière ? La Ligue des droits de l'homme- vous le savez, mais je le rappelle -a été créée pour défendre un innocent victime de l'antisémitisme et de la raison d'État, le capitaine Dreyfus. Elle a étendu d'emblée son action à la défense de tout citoyen victime d'une injustice ou d'une atteinte à ses droits. Dès le début du XXsiècle, seule, elle porta la justice sociale et le droit des travailleurs. Madame la Première ministre, ne l'oublions pas à la Libération, un tiers des membres du comité central de la LDH avaient disparu, assassinés, morts en déportation ou fusillés. Victor Basch, son président, fut assassiné en 1944 avec son épouse Ilona par la milice et les nazis. Tout au long du XXsiècle et jusqu'à nos jours, cette grande association exerça avec vigilance et humanisme le contrôle des excès des pouvoirs publics. Sans elle et d'autres vigies, l'autoritarisme nous guette. Il peut prendre le dessus. les mille personnalités qui ont déjà signé une tribune publiée ce jour dans, je le dis dignement, mais fermement : « Ne touchez pas à la Ligue des droits de l'homme ! » Je vous demande, madame la Première ministre, d'affirmer, sans ambiguïté, qu'aucune menace ne pèse sur elle. Je vous demande d'affirmer devant le Sénat que vous désavouez les propos de votre ministre de l'intérieur.

depuis plusieurs semaines, certains, à l'Assemblée nationale, au Sénat ou dans des interviews, dénoncent ce qu'ils appellent « une dérive autoritaire ». C'est une accusation tout aussi grave que mensongère. Notre État de droit et notre République reposent sur des libertés fondamentales. Ces libertés, nous les défendons et nous les défendrons. Les associations de défense des libertés publiques et des droits de l'homme mènent également ce combat, et je crois que personne ici ne peut contester sérieusement qu'elles ont, dans notre pays, la capacité de prendre position et de s'exprimer librement, pleinement et sans restriction. C'est indispensable, et nous veillerons à ce que cela demeure. Comme d'autres acteurs associatifs, la Ligue des droits de l'homme joue son rôle en observant, en critiquant et en exigeant des réponses des acteurs publics. Lorsque l'État est mis en cause, nous écoutons et nous le prenons en compte. Je souhaite, comme tous les membres du Gouvernement, que les associations de soutien aux droits de l'homme poursuivent leur action de vigie, d'ailleurs largement financée par l'État et les collectivités. Il n'est donc pas question de baisser par principe la subvention de telle ou telle association. Mais dialoguer avec ces structures sur leurs actions est aussi une responsabilité, dès lors qu'il s'agit de financement public. Madame la présidente Assassi, pour en revenir à la Ligue des droits de l'homme, je connais l'histoire de cette grande association. Pendant longtemps, l'histoire de l'émancipation républicaine et celle de la LDH se sont mêlées. L'universalisme était un terreau commun. Il y a toujours eu des débats exigeants, des confrontations parfois. Sans remonter à l'affaire Dreyfus, je pense à l'engagement de Madeleine Rebérioux ou de Me Henri Leclerc.

J'ai beaucoup de respect pour ce que la LDH a incarné, mais je ne comprends plus certaines de ses prises de position. Très bien ! Cette incompréhension n'est pas nouvelle. Elle s'est fait jour dans les ambiguïtés de cette association et elle s'est confortée depuis quelques mois. ! Je rappelle que cette association a attaqué un arrêté interdisant le transport d'armes par destination à Sainte-Soline.

Madame la présidente Assassi, la liberté d'expression et la liberté de manifester pacifiquement sont fondamentales en démocratie. Avec le Gouvernement, avec la grande majorité d'entre vous sur ces travées, je veux rendre hommage aux policiers et aux gendarmes, qui connaissent leur devoir d'exemplarité

La parole est à M. Didier Rambaud, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. et indépendants. Ma question s'adresse à M. le ministre délégué chargé des comptes publics. Qu'elles soient fiscales, sociales ou douanières, les fraudes sont une réalité persistante en France. Élément déterminant de notre contrat social, la lutte contre la fraude est un sujet préoccupant, un exemple de cause commune qui doit faire concorde. Dans un contexte où la maîtrise de nos finances publiques s'impose plus que jamais face aux crises que nous traversons, notre pays doit continuer de lutter contre toutes les fraudes. Depuis la loi du 28 octobre 2018

L'année 2022 est également une année significative. Les montants mis en recouvrement après contrôle fiscal ont atteint le niveau inédit de 14,6 milliards d'euros au total. Concernant la fraude au recouvrement social, le réseau des Urssaf a plus que doublé le montant des redressements réalisés depuis dix ans, lequel est passé de 320 millions d'euros en 2013 à 788 millions d'euros en 2022. Quant aux aux résultats de la douane, ils sont de nouveau historiques pour plusieurs segments de la fraude, comme les contrefaçons ou les trafics de tabacs. Ils devraient être accompagnés, je l'espère, d'un renforcement de nos outils dans la lutte contre la fraude douanière grâce au projet de en effet, des progrès peuvent indéniablement être réalisés. Il y a quatre mois, monsieur le ministre, nous débattions dans cet hémicycle de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. important travail de réflexion, associant les parlementaires de tous les groupes, a été engagé sur votre initiative, l'objectif étant d'aboutir à un plan d'action. Monsieur le ministre, que compte faire le Gouvernement pour continuer de renforcer notre lutte contre la fraude, sous toutes ses formes ?

je le dis solennellement devant vous, la lutte contre la fraude n'est pas qu'une question de deniers publics. C'est aussi, et probablement avant tout, une question de confiance dans l'action publique, de confiance de nos concitoyens, nos concitoyens, de cette classe moyenne qui a parfois le sentiment de payer trop parce que certains choisissent de ne rien payer du tout. La lutte contre la fraude est un enjeu autant de finances publiques que de cohésion nationale, et nous devons être implacables

Dans certains cas, on a l'impression qu'il n'y aurait que de la fraude fiscale et, dans d'autres, uniquement de la fraude sociale. Nous devons nous attaquer à toutes les fraudes, qu'elles soient fiscales, sociales ou douanières. Tel est l'objectif du groupe de travail que j'ai mis en place et qui réunit des représentants de la quasi-totalité des groupes politiques de l'Assemblée nationale et du Sénat. Nous nous sommes réunis à plusieurs reprises ces derniers mois. Nous avons beaucoup travaillé, et je présenterai dans les prochaines semaines un plan complet de lutte contre la fraude fiscale, sociale et douanière. Je précise que

À Saint-Brévin-les-Pins, le 22 mars, le maire a été victime d'un incendie volontaire perpétré par l'extrême droite intégriste et identitaire, qui s'oppose à l'emménagement du centre d'accueil pour demandeurs d'asile dans sa ville. À Bordeaux, le 23 mars, des identitaires, qui menacent de mort le maire depuis des mois, ont mis feu à la porte de sa mairie. Ce n'est pas vrai ! À Metz, le 5 avril, le chanteur Bilal Hassani a dû annuler un concert, après avoir reçu des menaces d'un collectif d'extrême droite Des groupuscules identitaires, comme Les Remparts à Lyon ou L'Oriflamme à Rennes, multiplient les intimidations et les attaques xénophobes et homophobes. Vous mentez ! Partout, on s'inquiète d'une résurgence des violences d'extrême droite. Le directeur général de la sécurité intérieure déclarait récemment que ces violences constituent la principale menace à laquelle nous sommes confrontés. sept des dix dernières tentatives d'attentats venaient de l'extrême droite. Madame la Première ministre, le mandat que les Français vous ont donné au soir du second tour de l'élection présidentielle, c'était d'être un rempart contre l'extrême droite.

pour anticiper et détecter la formation des groupuscules, qu'ils soient d'extrême droite ou d'extrême gauche, qui sont à l'origine de troubles à l'ordre public. Le ministère de l'intérieur fait preuve de la plus grande fermeté en la matière. Je vous rappelle que nous avons dissous une association d'extrême droite, les Zouaves Paris, dont

tous les outils pour lutter le plus efficacement possible contre tous ces séparatismes. La parole

dignes d'un régime autoritaire, l'alimentent. Vous banalisez dangereusement le mot « terrorisme », attaché à une mémoire si douloureuse dans notre pays, pour qualifier des adversaires politiques. Vous menacez de priver de subvention une association comme la Ligue des droits de l'homme, garante du respect de nos libertés publiques. Vous n'êtes pas le rempart contre l'extrême droite, vous êtes sa passerelle vers le pouvoir

Lors d'une étude de grande ampleur, l'Anses a trouvé 77 pesticides et résidus dans l'eau traitée. Parmi eux, le chlorothalonil a attiré l'attention des autorités, puisque ses métabolites ont été trouvés dans plus d'un prélèvement sur deux

Et pour cause : les filières de traitement conventionnelles ne parviennent pas à se débarrasser de ce fongicide. Les technologies pour lutter contre ce métabolite sont à la fois coûteuses et énergivores. Ce fongicide, longtemps utilisé dans de nombreuses cultures, est considéré comme un cancérogène probable depuis 2006. est interdit en Europe depuis 2019. Pourtant, alors que l'on sait que certains résidus de pesticides peuvent être présents dans l'environnement plusieurs années après leur interdiction, le chlorothalonil n'avait jamais été recherché dans notre eau potable. Alors que l'on sait que la molécule provoque des tumeurs rénales chez les souris, les recherches sur la santé humaine demeurent lacunaires. Or celles-ci pourraient justement permettre de rassurer la population, voire, si c'est justifié, d'abaisser le niveau d'exigence sanitaire. Sur un sujet aussi sensible que l'accès à l'eau potable, dans le contexte de tensions croissantes que nous connaissons sur le partage de la ressource, il nous faut des éléments de réponse précis et des solutions nationales à court et à long terme, sous peine d'aboutir à une fracture de confiance, mais aussi à une fracture territoriale, avec de petits réseaux

j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet hier à l'Assemblée nationale. Je vous remercie de me donner l'occasion de le redire aujourd'hui devant le Sénat : l'eau est notre bien le plus précieux, et le Gouvernement met évidemment tout en oeuvre pour en assurer et surveiller la qualité. Il s'agit d'un enjeu majeur de santé publique. La surveillance de la qualité de l'eau est une préoccupation quotidienne. C'est bien pour cette raison que, sous l'autorité du ministère de la santé et de la prévention, la direction générale de la santé missionne régulièrement les agences d'expertise françaises pour disposer de connaissances sanitaires sur les pesticides et leurs métabolites. Le but de ces campagnes exploratoires est de disposer des données les plus précises possible pour évaluer les risques sanitaires. L'Anses, vous l'avez dit, a publié la semaine dernière les principaux résultats de la dernière campagne exploratoire 2020-2022, relative aux polluants émergeant dans l'eau potable. Ce rapport met en évidence une contamination des ressources en eau destinées à la consommation humaine en France métropolitaine par différents métabolites, dont le chlorothalonil, un fongicide interdit en France depuis 2020. À ce jour, la campagne exploratoire de l'Anses a mis en évidence des concentrations maximales de 2 microgrammes par litre, la valeur sanitaire transitoire permettant de prévenir d'un risque sanitaire est de 3 microgrammes par litre. Les échantillons prélevés ne présentent donc pas de risque sanitaire à ce stade. Plusieurs responsables de la production et de la distribution d'eau ont déjà intégré le chlorothalonil et ses métabolites dans leurs plans de surveillance. Le programme de contrôle des agences régionales de santé va progressivement intégrer, à partir de 2023, le chlorothalonil et ses métabolites dans le contrôle sanitaire des eaux pour rendre des résultats fiables. Ces éléments permettent de poursuivre le travail d'amélioration de la qualité des eaux, en particulier dans les zones de captage, et d'adapter et de différencier nos mesures en fonction des spécificités territoriales, comme l'a annoncé le Président de la République lors de la présentation du plan Eau le 30 mars dernier. Vous le voyez, le Gouvernement est pleinement mobilisé. Il suit ce sujet essentiel avec une grande vigilance,

la crédibilité de votre politique en matière de pesticides et de qualité de l'eau s'effrite de jour en jour. Que répondez-vous à la population inquiète de boire de l'eau du robinet ? Que répondez-vous aux collectivités qui s'interrogent sur les coûts de dépollution ?

Aujourd'hui, quand on fait le bilan, très peu de choses ont avancé. Les pesticides sont toujours dans la place, sur le sol, dans l'eau et dans l'air. L'agriculture biologique reste un parent pauvre, et cela malgré la succession des ministres de l'agriculture. Je me dis avec dépit

Vanina Paoli-Gagin, pour le groupe Les Indépendants - République et Territoires. Dans nos villes comme dans nos campagnes, ces édifices sont un trait saillant du visage de la France, et ils contribuent à sa tenue et à son rayonnement. Nous avons le devoir de préserver ces richesses héritées, pour les transmettre aux générations futures, lesquelles, à leur tour, en seront responsables.

Face aux défis protéiformes de la préservation patrimoniale, dont l'ampleur ne cesse d'enfler, les communes peinent à conserver et à valoriser ces trésors. Elles rencontrent également des difficultés à les assurer, madame la ministre, car le secteur privé n'a pas développé les réponses idoines. Les élus locaux, notamment nos maires, se sentent démunis. Il est urgent d'engager une vaste réflexion sur la préservation du patrimoine communal et la capacité de l'assurer.

immobilier. Il viendrait utilement compléter celui qui a été proposé récemment par M. Stéphane Bern et il permettrait de mobiliser concrètement l'État aux côtés des communes, en faveur de ce patrimoine qui ne relève pas de sa compétence. Nous devons, ensemble, relever le défi de la préservation de ce patrimoine remarquable

Après le rachat par l'américain Heico de l'entreprise Exxelia, fleuron français de l'électronique, c'est à présent la PME Segault qui menace de passer sous pavillon américain. Pour ceux d'entre vous qui ne la connaissent pas, mes chers collègues, je rappelle que cette PME fabrique, entre autres, les pièces de robinetterie de haute technologie qui équipent nos centrales nucléaires et les chaufferies de nos sous-marins nucléaires, ou encore celles de notre porte-avions Charles-de-Gaulle- c'est pourquoi j'associe à ma question Indispensable au nucléaire civil comme militaire, Segault entre, à double titre, dans le champ des secteurs stratégiques visés par la réglementation sur le contrôle des investissements étrangers. Si nous ne pouvons pas envisager que cette entreprise passe sous contrôle américain, monsieur le ministre, c'est parce que le Patriot Act permet au Gouvernement américain de demander l'accès à tout type d'information détenue par une entreprise américaine, quelle que soit sa localisation dans le monde et sans aucune justification. Ainsi, dans le champ de compétences de Segault, des informations, même partielles, sur la conception de nos infrastructures nucléaires pourraient être transmises sans obstacle juridique. Il y a donc un double enjeu, de souveraineté

Quels outils juridiques et quels moyens financiers allez-vous mobiliser pour que Segault revienne durablement dans le giron français ? Allez-vous activer, monsieur le ministre, le décret de 2014 relatif au contrôle des investissements étrangers ? Allez-vous chercher des acquéreurs nationaux ?

Bien sûr, nous sommes particulièrement vigilants, parce que Segault est une entreprise stratégique et parce que les États-Unis, comme vous l'avez rappelé, disposent d'une réglementation particulièrement offensive, qui pourrait menacer la confidentialité et la souveraineté des informations relatives aux technologies développées par Segault.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le 8 janvier 1964- il y aura bientôt soixante ans -le général de Gaulle, en conseil des ministres, déclarait : « La Chine est là. Vivre comme si elle n'existait pas, c'est être aveugle Le 27 janvier suivant, la reconnaissance par la France de la République populaire de Chine était annoncée, dans un environnement international pas forcément plus conciliant que celui que nous connaissons aujourd'hui. Quelle vision ! Le Président de la République rentre de Chine. Nous approuvons ce voyage, qui nous confirme que, finalement, la Chine garde son cap, en fonction de ses seuls intérêts stratégiques. Dès lors, monsieur le ministre, pourquoi cette déclaration à l'emporte-pièce sur Taïwan ? Entre Europe, Chine et États-Unis, quelle est la stratégie française ?

vous l'avez rappelé, le Président de la République a effectué une visite d'État en Chine du 5 au 8 avril dernier. Il était accompagné par la présidente de la Commission européenne. Cette visite avait plusieurs objectifs. D'une part, il s'agissait de relancer la relation, en particulier dans le domaine des échanges humains. À ce titre, des accords ont été conclus dans le domaine du développement durable, de la coopération culturelle et de l'économie agroalimentaire et aéronautique. Nous avons lu le journal ! D'autre part, l'enjeu était d'avoir un dialogue franc sur l'Ukraine. République a fait valoir les positions européennes, a appelé la Chine à s'engager dans la recherche d'une solution et a alerté son homologue chinois sur les conséquences que tout soutien militaire à la Russie aurait sur la relation entre Union européenne et Chine. Des points de convergence sont ainsi apparus l'opposition à l'emploi de l'arme nucléaire, le respect du droit international humanitaire et la nécessité de trouver une issue au conflit sur la base du droit international. Et Taïwan ? Un autre enjeu de ce déplacement était de marquer notre unité européenne. La présence de la présidente de la Commission était un point essentiel pour le Président de la République, qui tenait à montrer

La France qui, je le crois, est fermement attachée au droit, à la liberté de navigation et à l'avenir de l'Indopacifique ne peut rester étrangère à la montée des tensions autour de Taïwan, où les incursions militaires chinoises sont de plus en plus fréquentes et structurées.

nos partenaires de l'Union européenne le sont encore moins. Une tentative d'action de vive force sur Taïwan par la Chine, comme celle qui a été perpétrée en Ukraine par la Russie, n'est plus à exclure. L'Armée populaire s'y prépare au quotidien. Nous devons donc rester extrêmement prudents dans toutes nos déclarations.

comme vous le savez, de délai représente un seuil critique, au-delà duquel la perte de chance est réelle. À l'inquiétude des patients s'ajoutent les alertes des professionnels du soin. Les pompiers volontaires nous disent ainsi que la longueur des trajets risque non seulement de rendre risque non seulement de rendre les employeurs réticents à laisser leurs salariés s'engager, mais aussi de dissuader les volontaires eux-mêmes. Cette situation n'est pas isolée. Les risques de fermetures de services d'urgences ou de maternités se multiplient

Autoriserez-vous cette organisation, monsieur le ministre, afin de maintenir le service ouvert le temps de trouver d'autres solutions ? Concernant les intérimaires, allez-vous rétablir l'équité de traitement entre établissements publics et privés ? Il est clair que le Ségur n'a pas suffi à redonner de l'attractivité aux carrières médicales hospitalières ... Monsieur le ministre, Monsieur le ministre, allez-vous enfin proposer une réforme d'ampleur pour revaloriser les salaires et améliorer les conditions de travail à l'hôpital ? Ou attendrez-vous qu'il y ait encore dix, cinquante ou cent fermetures, comme à Feurs ?

notamment dans les pays extraeuropéens, en particulier pour nos marchés en Afrique du Nord et de l'Ouest. Or l'Anses a décidé, de façon unilatérale, de ne plus permettre l'usage de la phosphine, qui reste pourtant homologuée, Paradoxalement, les céréales importées en France continueront, elles, à être traitées à la phosphine. En effet, aucune réglementation européenne n'interdit l'utilisation de cet insecticide. C'est un non-sens total Comment l'Anses a-t-elle pu édicter une telle règle sans concertation ? A-t-on bien mesuré les conséquences de cette interdiction ? Cette sentence est également dramatique pour les pays du bassin méditerranéen qui dépendent de la France et dont la sécurité alimentaire est menacée par cette décision absurde. Aussi, monsieur le ministre, j'aimerais connaître les solutions que le Gouvernement peut proposer pour préserver nos exportations de céréales et empêcher les crises alimentaires dans les pays qui dépendent de nos exportations.

C'est celui de la sécurité alimentaire mondiale.

Cette modification, présentée comme technique à l'origine, aboutit en effet à les priver de la récupération de la TVA sur des travaux lourds dits « d'agencement et d'aménagement de terrains », ce qui exclut nombre de chantiers, comme des terrains de football, des aires de jeu ou encore des pistes cyclables. Surtout, cette réglementation comporte des éléments de complexité supplémentaires, avec, au sein d'un même projet, des dépenses qui restent éligibles et d'autres qui ne le sont plus, alors qu'un projet est un tout. Aussi, ma première question est simple : envisagez-vous de revenir sur cette réglementation très mal vécue par les collectivités locales ou, à tout le moins, d'intégrer la part de TVA dans l'assiette subventionnable ?

Mizzon, vous avez raison, l'automatisation du FCTVA conduit à une redéfinition de l'assiette des dépenses ouvrant droit à compensation. Dans la collecte des données comptables nécessaires au calcul automatique des attributions, certaines dépenses ont été exclues de l'assiette. des dépenses engagées par les collectivités, telles que celles que vous avez citées. D'autres dépenses qui n'étaient pas éligibles le sont désormais. C'est le cas, par exemple, des investissements réalisés par des collectivités pour des biens immobiliers qu'elles mettent à la disposition de tiers.

constitue une mesure favorable aux collectivités, puisqu'elle permet la disparition du non-recours, qui concernait jusqu'à présent les plus petites d'entre elles. Pour autant, une évaluation sera conduite à la mi-2023. La question des dépenses d'aménagement de terrain sera examinée de très près, monsieur le sénateur, dans la suite des débats que nous avons menés sur le projet

construire 5 000 équipements sportifs un jour et, le lendemain, sortir de la dépense éligible les dépenses qui les financent.

La parole est à M. François Bonhomme, pour le groupe Les Républicains.

droit fondamental s'il en est. Il y a, dans cette instrumentalisation systématique du droit, une dérive qui interroge. Comment l'État peut-il soutenir et subventionner des associations faisant profession de jeter l'opprobre sur les forces de l'ordre,

Pays-Bas. Permettez-moi de rappeler le contexte de la prise de parole du ministre, que vous avez interrogé, dans le cadre d'une audition en commission, sur la possibilité de supprimer les subventions versées à cette association. La Ligue des droits de l'homme est une association ancienne et respectable, dont le nom a été associé, c'est vrai, à des combats qui font honneur à la République. Pour autant, certaines de ses prises de position récentes interrogent, et ce n'est pas lui faire injure que de le reconnaître. Je citerai par exemple son absence au procès des attentats de en 2020, ou encore sa décision, difficile à comprendre, de défendre

et de 233 000 euros des collectivités territoriales. Il est donc légitime que l'État s'assure que les actions conduites par une association bénéficiant de financements publics sont en phase avec l'objectif qu'elle déclare, ainsi qu'avec nos valeurs républicaines.

pour éviter le pire. Ils espéraient que le Président de la République saurait en tenir compte. Or, en retour, après onze journées de très forte mobilisation dans une grande responsabilité intersyndicale, il reste sourd. Comme lui, votre gouvernement prend une attitude arrogante. Votre autosatisfaction montre combien vous êtes déconnectée des réalités que vivent nos concitoyens. Vous méprisez l'intersyndicale, unie contre cette réforme. Vous méprisez l'opposition parlementaire, notamment au Sénat, en utilisant tous les artifices, afin de brider le débat. Vous méprisez les millions de Françaises et de Français qui manifestent leur opposition depuis des mois dans la rue, et cela malgré l'inflation qui grève le budget de leur Face à la colère qui s'exprime, vous restez insensible aux revendications légitimes. Ainsi, vous affaiblissez nos institutions, notre démocratie et notre modèle social. Cette réforme laissera des séquelles profondes dans notre pays. Ces dernières semaines, vous avez usé de tous les stratagèmes, jusqu'aux magazines, pour faire diversion et tenter de tourner la page de cette séquence. Mais les Français ne sont pas dupes ils n'oublieront pas. Votre réforme est inutile et injuste, c'est une régression sociale. Madame la Première ministre, vous êtes dans l'impasse. Comment entendez-vous gouverner après avoir méprisé à ce point les corps intermédiaires ? Comment entendez-vous apaiser les tensions et renouer le dialogue social ? Je ne vois qu'une issue : le retrait

les zones blanches médicales concernent tous les territoires, et les aides financières ponctuelles ne permettent pas, à elles seules, d'attirer les jeunes médecins. Le Sénat a adopté l'an dernier

dans les zones caractérisées par des difficultés d'accès aux soins. Chaque année, près de 4 000 internes auraient ainsi été déployés dans les zones sous-dotées. L'article 37 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 prévoit un dispositif analogue. Les étudiants resteraient dans la région où ils ont suivi leurs études et bénéficieraient d'une rémunération adaptée. Monsieur le ministre, vous avez confié à des personnalités qualifiées une mission sur la refonte du troisième cycle de médecine générale. Pouvez-vous nous faire part de leurs conclusions et nous préciser la date d'entrée en vigueur de l'article 37 de la loi

pour les étudiants de troisième cycle de médecine générale d'effectuer un stage d'au moins six mois en médecine ambulatoire. Cette mesure n'a jamais été mise en place. Tout en regrettant le temps perdu, nous nous réjouissons que le Sénat ait enfin été entendu. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour le groupe Les Républicains.

Si le rapport évoque le progrès des connaissances scientifiques et médicales, il dresse un constat, que certains qualifient de sévère, sur une certaine inefficacité des plans Chlordécone qui se sont succédé, inefficacité qui explique le sentiment de défiance et de colère des Antillais. Sa conclusion est, hélas, d'actualité : ce qui est arrivé aux Antilles doit servir de modèle à l'État pour gérer les pollutions que nous ne manquerons pas de découvrir ; une vision à long terme s'appuyant sur la recherche et associant tous les acteurs est dorénavant nécessaire.

ma question est simple. Avez-vous mis au point une stratégie permettant de faire face à ces contaminations, une stratégie qui soit réfléchie et qui englobe les aspects sanitaires, économiques, environnementaux et sociaux ? Comment comptez-vous associer et informer clairement la population pour éviter le contre-modèle du chlordécone

je vous rappelle que, depuis un peu plus de deux ans, un site internet, InfoSols, certes méconnu de la plupart de nos concitoyens, géré par le ministère de la transition écologique, recense toutes les pollutions existantes. Et il est mis à jour de manière régulière.

Un plan d'action dévoilé en janvier dernier par mon ministère a mis l'accent sur la nécessité de connaître l'existant, de recenser et d'améliorer les informations ou encore de mesurer les endroits où il y a potentiellement des problèmes pour la santé. Là aussi,

de l'intelligence artificielle générative ». Je vous rappelle que, dans ce débat, le Gouvernement aura la faculté, s'il le juge nécessaire, de prendre la parole immédiatement après chaque orateur pour une durée de deux minutes ; l'orateur disposera alors à son tour du droit de répartie, pour une minute.

capacités de calcul et de stockage des données. C'est un sujet hautement complexe, car expliquer ce qu'est un système neuronal artificiel n'est pas chose aisée. L'idée est de copier le modèle de fonctionnement du cerveau humain.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, « l'intelligence artificielle générative, une technologie capable de créer de nouveaux contenus, écrits ou images, recèle un fort potentiel, et ses impacts sociaux sont multiples. Dans le champ économique, l'intelligence artificielle générative, en permettant l'automatisation de certaines tâches répétitives et sans grande valeur ajoutée, accroît l'efficacité du travail et donc sa rentabilité. En créant de nouveaux produits ou services basés sur cette technologie, elle est potentiellement créatrice d'emplois. « Toutes ces potentialités peuvent néanmoins être disruptives pour notre modèle économique actuel. En générant un risque de destruction d'emplois ou en limitant la nécessité d'acquérir de nouveaux savoirs, l'intelligence artificielle générative obligera plusieurs secteurs industriels à s'adapter pour demeurer compétitifs. « Les risques politiques et éthiques existent aussi pour nos valeurs démocratiques, notamment par la génération de faux contenus, qu'ils soient écrits, visuels ou sonores, qui viendraient nourrir propagandes diverses et désinformation. Les répercussions sur les processus électoraux sont possibles. À mesure que les intelligences artificielles génératives se perfectionneront, il deviendra de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux. Ce que vous venez d'entendre, mes chers collègues, ce n'est pas un discours rédigé exclusivement par mes soins ou par ceux de ma collaboratrice. Ce début d'intervention a été généré à près de 95 % par l'application ChatGPT. Monsieur le ministre, vous avez qualifié ChatGPT de « perroquet approximatif Utilisé dans le contexte précis d'une intervention dans l'hémicycle, le trouvez-vous convaincant ou maintenez-vous votre jugement ? « Distinguer le vrai du faux », « création d'emplois » et « potentiel disruptif En une minute, je pense que vous avez pu relever les principaux apports et risques de l'intelligence artificielle générative, limites et promesses dont la machine elle-même semble parfaitement consciente. Vous constatez également la nécessité qui est la nôtre de les identifier pour combler le vide juridique entourant le développement de cette technologie, dont on ne peut nier le potentiel de fascination et qui évolue à une vitesse sidérante. Comme toute innovation majeure dans l'histoire de l'humanité, les intelligences artificielles génératives font planer le spectre de destructions d'emplois, d'un remplacement de la force humaine par l'agilité de la machine et d'une forme de simplification de l'organisation du travail par la suppression du facteur humain. On oublie seulement de dire que les nouvelles technologies, quelles qu'elles soient, créent souvent davantage d'emplois qu'elles n'en détruisent. Par ailleurs, leur développement ne signifie pas systématiquement un abandon des savoir-faire antérieurs. L'intelligence artificielle peut au contraire permettre la création et l'acquisition de nouvelles compétences. Le secteur qui sera le plus directement affecté par leur développement sera sans surprise celui de l'informatique. Cela induira nécessairement une adaptation et, par là même, une expertise plus poussée de la part des ingénieurs, ainsi que la création de nouveaux métiers attractifs. L'une des principales craintes généralement partagées face à un tel potentiel est aussi de voir l'humain dépassé par sa créature. Toutefois, cette source d'intelligence repose encore et toujours sur l'humain, tandis que les intelligences artificielles génératives ne demeurent, en tout cas en 2023, que des fabriques d'illusions. En dépit de leur qualité, le contenu proposé ne se fonde que sur des corrélations statistiques, un volume de données certes exponentiel, mais toujours limité. Sans l'humain, point de machine, Ces inventions posent néanmoins de réelles questions éthiques et philosophiques. Comme toutes les technologies qui les ont précédées, par exemple internet, elles sont un, à la fois poison et remède selon l'usage que l'on en fait. Bien sûr, entre de mauvaises mains, ces outils sont dangereux, parce qu'ils sont hautement capables de tromper notre vigilance ou d'être utilisés pour défendre des intérêts particuliers. Mais cette créature-là ne nous échappera que si nous ne nous ne nous posons pas les bonnes questions et si nous n'anticipons pas ses effets pervers. Les mêmes interrogations relatives à la régulation, aux normes et à une éventuelle gouvernance mondiale se posent aujourd'hui pour l'intelligence artificielle, comme elles se posent depuis plus de vingt-cinq ans face à l'essor d'internet. Force est de constater que nous avons appris en marchant. Il pouvait difficilement en être autrement, faute de précédent. Toutefois, nous disposons aujourd'hui de cette expérience, d'un corpus de réflexions, de normes et d'une jurisprudence- tout cela peut nous guider. faut nous servir de ce savoir empirique. Une difficulté demeure cependant : face à une technologie par nature dynamique, qui progresse sans cesse, le risque de caducité rapide des normes définies à un moment précis est réel. Il nous faut donc être plus rapides que la machine. Et c'est je pense, que se situe l'aspect le plus positif de cette technologie novatrice : en nous débarrassant du superflu, elle peut aussi nous permettre de nous concentrer sur l'essentiel. En vérité, elle nous lance un défi : elle nous invite à un regain d'intelligence. d'intelligence. Si l'IA générative peut nous affranchir de certaines tâches répétitives, doit-elle fatalement nous rendre intellectuellement paresseux ? C'est à l'humain de montrer qu'aucune machine ne peut surpasser son intelligence, son jugement, son esprit critique et sa remarquable capacité d'adaptation. Qu'ils soient positifs ou négatifs, les impacts sociaux et économiques de l'intelligence artificielle générative doivent être évalués. Nous ne pourrons pas faire l'économie d'une réflexion éthique, afin que cette technique puisse être utilisée au bénéfice de l'intérêt général. » Cette conclusion, mes chers collègues, m'a été proposée par l'application ChatGPT ... Je vous laisse apprécier sa pertinence Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la révolution numérique a suscité un véritable bouleversement du monde du travail, opérant une transformation en profondeur de notre modèle économique et des métiers qui en constituent l'architecture. Il est estimé qu'environ la moitié des métiers que les jeunes écoliers d'aujourd'hui exerceront demain n'existent pas encore.

Nous sommes aujourd'hui dans un système où l'utilisateur est poussé par un ensemble de plateformes et de systèmes algorithmiques à générer toujours plus de données, au service finalement d'annonceurs, de publicitaires et de producteurs d'intelligence artificielle.

Parce que « mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde », comme disait Albert Camus, il convient de rappeler que l'intelligence artificielle n'est ni artificielle ni intelligente. Considérer le logiciel ChatGPT comme intelligent, c'est se tromper lourdement sur la nature de notre débat et sur ses enjeux écologiques, politiques et sociaux. ChatGPT n'est pas simplement un automate computationnel. Il implique l'exploitation des ressources minérales- terres rares -et humaines nécessaires à sa production et à son fonctionnement. Il dépend du travail gratuit des millions d'utilisateurs dont les requêtes améliorent l'algorithme. ces « micro-tâches », rémunérées moins de 2 euros de l'heure, on s'affranchit du salariat et on précarise, à l'heure actuelle, des centaines de milliers de personnes à travers le monde, selon les travaux d'Antonio Casilli. Comme toute révolution technologique, la révolution numérique est au coeur d'un affrontement de classes ; l'industrie du numérique a pour seule obsession de casser le coût du travail, en espérant substituer du capital mort au capital vivant. Pourtant, cette révolution numérique pourrait créer de nouveaux métiers, augmenter les besoins en formation initiale et professionnelle et offrir la possibilité de réduire le temps de travail pour gagner du temps libre. Néanmoins, l'orientation choisie par l'industrie du numérique, avec la collaboration aveugle de nos gouvernants, est manifeste il s'agit d'exercer une pression sur les salaires et sur l'emploi, en captant la valeur, plutôt que d'améliorer l'efficacité sociale du travail. Il s'agit aussi de transformer en plateformes nos services publics et administratifs, créant davantage d'insécurité sociale. Cette industrie est dominée, à l'exception de la Chine, par une poignée de firmes américaines concentrant des capitalisations boursières démesurées et motivées par une visée politique mondiale, celle d'un capitalisme à son paroxysme, où l'on peut s'arroger certaines prérogatives étatiques en toute impunité. Face à cela, la France et l'Union européenne ont joué le jeu de la en reléguant le choix de l'outil numérique ou d'un prestataire technique à une logique utilitariste, sans prendre en compte les aspects politiques et stratégiques. Il est impératif de reprendre la main sur notre destin et de choisir la société dans laquelle nous voulons vivre demain. Nous devons nous réapproprier collectivement nos données sous forme de communs, en exigeant la transparence et la lisibilité des algorithmes participant à l'apprentissage automatique. Cet espoir de transition numérique, je le place aussi dans notre jeunesse, dans ce nombre considérable de jeunes adultes qui ne supportent plus de faire des « jobs à la con entendez par là, mes chers collègues, un travail auquel on ne trouve pas de sens, qui prive d'une réelle protection sociale et dans lequel règne une hiérarchie autre que celle de la compétence. Parmi ces jeunes, nombreux sont ceux qui veulent créer et entreprendre, mais pas forcément en fondant une start-up pour la revendre au plus offrant et faire fortune. Leur objectif est plutôt d'entretenir et de rendre accessibles, un réseau numérique, des communs mondiaux d'innovation partagée. Cette jeunesse pense nouveaux modes de production, coopératives, économie sociale et solidaire, économie circulaire, lutte contre l'obsolescence programmée et mise en commun Ces nouveaux terrains de la lutte de classe, où l'on prépare une alternative au monde numérique capitalistique tel qu'il est conçu aujourd'hui, on les retrouve dans les ateliers coopératifs de fabrication et de création numériques, au sein des communautés de développement de logiciels libres, mais aussi dans les plateformes numériques coopératives. Ces tiers lieux préfigurent une possible République des communs. Oui, mes chers collègues, cette révolution numérique, à l'oeuvre depuis des années déjà, nous place au pied du mur du dépassement de la condition salariale. Mais aujourd'hui, nous devons choisir

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le développement exponentiel de la technologie signifie-t-il la fin programmée de l'humanité, telle que nous la connaissons ?

sur nos modèles sociaux, politiques et démocratiques, notamment par de possibles abus en matière de désinformation, de manipulation des opinions ou de contrôle des individus. Si la presse se fait, jour après jour, l'écho des nouvelles prouesses de ChatGPT, des pays comme l'Italie ou le Canada l'ont interdit, tout comme d'autres ont banni TikTok. sur l'intelligence artificielle, comme l'ont demandé Elon Musk et un millier de scientifiques ? Peut-être, mais ne soyons pas dupes : au-delà des considérations éthiques, il y a là pour le dirigeant de SpaceX et de Twitter une occasion de régler ses comptes avec OpenAI dans la course effrénée à laquelle se livrent les entreprises pour la captation du marché. Faut-il de la régulation et une intervention des pouvoirs publics pour mieux encadrer ces futures applications ? Assurément. Je le demande depuis dix ans, rapport après rapport, car je mesure la puissance transformatrice des nouvelles technologies, mais aussi leurs effets incertains et potentiellement dangereux sur la mise en réseau du monde.

et coauteure à ce titre d'une proposition de résolution européenne, je veux en souligner le caractère précurseur, l'Europe étant la première à se doter d'un cadre juridique en la matière. Cependant, si son approche par le risque est pertinente, cette proposition de règlement ne résout pas, hélas, les questions éthiques que posent les algorithmes gourmands de nos données données et les modèles économiques qui les sous-tendent. Comme je le réclamais pour le DSA, il faut exiger la transparence absolue, des audits indépendants et, tant avant la mise sur le marché d'une application ou d'un logiciel que tout au long de leur cycle de vie,

Or par manque de stratégie industrielle ces dernières années, l'Europe a été largement distancée par les États-Unis et la Chine, car ces États ont massivement investi dans la recherche et le développement de leurs propres entreprises, qui dominent aujourd'hui le monde. Si l'Europe ne veut pas totalement disparaître de la carte des technologies de demain, monsieur le ministre, elle doit se réveiller et sortir de ces dépendances dangereuses. Avec l', les États-Unis vont investir près de 348 milliards de

décider de notre avenir, ainsi qu'un investissement dans la recherche et un soutien assumé à notre écosystème européen, grâce à un : tel est le triptyque pour lequel je ne cesse de plaider. La maîtrise des technologies les plus avancées est devenue un enjeu géopolitique. Cette approche n'est donc pas du protectionnisme ; c'est la seule manière de promouvoir un monde valeurs fondamentales, un monde qui n'exprime ni le modèle de la- le profit avant la sécurité -ni le modèle du contrôle social par le parti communiste chinois. L'Europe doit aussi peser dans les instances mondiales où s'élaborent les protocoles et les standards.

en faveur d'une intelligence artificielle qui soit au service de l'humain, fiable et éthique. Il y a là un enjeu de civilisation. La parole

À l'heure où 100 millions de personnes ont les yeux rivés sur leur écran pour admirer les prouesses aussi extraordinaires qu'effrayantes du robot ChatGPT, la société semble programmée pour une forme d'obsolescence de ses modes de production et d'éducation.

technologie- car nous n'en sommes qu'aux balbutiements -dépassent déjà les performances de tous les outils que nous connaissions jusqu'ici. Les équilibres économiques du monde vont être bouleversés, et Google pourrait être remisé au rang de curiosité du passé. Alors que la parole publique et les fonctions électives sont plus que jamais remises en question dans notre pays, le peuple va chercher les réponses à ses questions auprès d'algorithmes pré-entraînés dont la capacité stupéfiante à singer l'intelligence humaine crée les conditions d'une dystopie nouvelle. Les craintes que nous que nous entrevoyons avec une telle technologie ne font que rappeler l'intrusion du numérique dans nos vies depuis de nombreuses années. Nous assistons à l'extension de l'ubérisation au domaine de la pensée. Cela pose la question de la liberté et du rapport à la réalité. Créées dans la Silicon Valley, ces ces technologies diffusent un conformisme idéologique fidèle au progressisme de ses concepteurs et aux références anglo-saxonnes. C'est donc l'esprit critique et notre souveraineté qui sont menacés. L'intelligence artificielle générative représente aussi une occasion de développer le secteur de la santé et de refondre l'éducation nationale en un système d'instruction tourné vers l'innovation et l'ingénierie. Le monde accélère. Monsieur le ministre, en marche ! Aussi, qu'avez-vous prévu pour promouvoir le développement des entreprises françaises dans ce domaine et réfléchir aux limites éthiques que nous devons mettre en place pour empêcher l'effondrement de notre pays et assurer notre compétitivité ?

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, de ChatGPT à Midjourney en passant par DeepMind, l'intelligence artificielle a franchi des étapes inimaginables il y a encore quelques années, une évolution qui suscite à la fois intérêt et intérêt et inquiétudes. Intérêt, car l'intelligence artificielle dite « générative »- celle qui nous intéresse aujourd'hui -est une nouvelle révolution industrielle, porteuse d'innovations à venir tant pour les biens que pour les services. Inquiétudes, car son mode de fonctionnement est de prendre

Nous n'en sommes pas là, heureusement, mais n'attendons pas que certains des enjeux de l'intelligence artificielle soient hors de contrôle. Au moment où nous parlons, je ne pense pas que la question soit encore celle de savoir si cette technologie est souhaitable ou non. Elle est déjà à l'oeuvre, et les investisseurs s'y engouffrent avec allégresse. Par conséquent, nous en sommes plutôt à savoir comment l'encadrer, afin de ne pas la subir. L'éthique est un des premiers enjeux de l'intelligence artificielle générative. Par exemple, doit-on permettre ses usages pour des prescriptions médicales, des fonctions d'encadrement du travail, ou encore des programmes de surveillance ? Ce dernier point me conduit à celui de la protection des données personnelles. Tout d'abord, on doit se réjouir que deux plaintes aient été récemment déposées en France auprès de la

À une autre échelle que celle des pays, on observe également que des institutions se mobilisent. Je pense par exemple à l'interdiction par Sciences Po d'utiliser le robot conversationnel d'OpenAI en dehors d'un encadrement pédagogique.

Une vaste réflexion menée au sein de l'éducation nationale pourrait permettre d'en circonscrire l'usage, au moins durant le temps scolaire. Il faut en tout cas rapidement s'intéresser à cet enjeu. Le RDSE, attaché à l'esprit des Lumières, souhaite que la question des sources soit également bien appréhendée vis-à-vis de cette technologie, qui peut alimenter contre-vérités et mauvaises informations.

Il faut en tout cas se préparer à une évolution des emplois, le plus important étant d'éviter leur précarisation, cette ubérisation que l'on a pu regretter dans certains secteurs. Aussi, monsieur le ministre, il revient à la puissance publique de s'engager fermement sur ce chantier, afin de rappeler que tout n'est pas permis à l'intelligence artificielle et que sa vocation devrait être de supprimer des tâches et non des métiers. En attendant, le groupe RDSE ne souhaite pas verser dans la technophobie, sous réserve que l'humanisme reste la valeur centrale du progrès.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis quelques mois, les intelligences artificielles sont au centre de l'actualité. Qu'il s'agisse de logiciels conversationnels tels que ChatGPT ou Eliza, de modèles de génération d'images et de vidéos, ou encore d'auto-encodeurs, pas une semaine ne passe sans que l'on mette à la une les prouesses de ces nouvelles technologies pouvant produire des contenus de manière autonome, suscitant tour à tour admiration et inquiétudes. En réalité, la très probable révolution industrielle que représentent les intelligences artificielles s'est amorcée il y a plusieurs années déjà. Nous en utilisons chaque jour sans le savoir. Au fil des mises à jour et de la collecte toujours plus massive de données, elles ne cessent de se perfectionner. Si elles partagent des similitudes avec les intelligences artificielles plus traditionnelles, les IA génératives soulèvent des problèmes spécifiques, notamment en matière d'éthique, de désinformation, de protection des données, ou encore de productivité et d'impact sur les emplois. Bien que des améliorations soient encore nécessaires pour qu'elles soient utilisables à une échelle industrielle, de nombreuses études montrent que leur éventuelle généralisation aura des impacts d'une ampleur inédite depuis l'arrivée de l'ordinateur. Ainsi, une étude menée par OpenAI, Open Research et l'université de Pennsylvanie avance que 80 % de la main-d'oeuvre américaine pourraient voir au moins 10 % de leurs tâches réalisées par une intelligence artificielle générative. Pour 19 % des travailleurs, 50 % de leurs tâches pourraient être prises en charge par ces nouvelles technologies, en particulier dans les domaines des services administratifs et juridiques, du management, des services financiers, du marketing, de la communication, ou encore du graphisme et de la conception. D'après une autre étude de la banque Goldman Sachs, 300 millions d'emplois pourraient à terme être menacés, mais la productivité au travail pourrait progresser de 1,5 point chaque année pendant dix ans, tandis que la hausse annuelle du PIB mondial pourrait atteindre 7 %, contre 2,9 % prévus pour 2023 par le FMI. Sans qu'il puisse être affirmé que certains métiers disparaîtront inévitablement, puisqu'un gain de productivité n'entraîne pas nécessairement la disparition d'un emploi, il est certain que le marché du travail sera bouleversé. De même, de nouveaux métiers apparaîtront et compenseront probablement le nombre de postes supprimés. Si une étude du Forum économique mondial estime que 87 millions d'emplois seront remplacés par des intelligences artificielles, elle met en exergue que celles-ci permettront la création de 95 millions d'emplois. Bien sûr, il ne s'agit à ce stade que de prévisions ; les effets de ces technologies sur le marché du travail devront de toute évidence être suivis de près, afin que nous puissions nous adapter à des conséquences imprévues de leur usage. En outre, si la France veut profiter pleinement des externalités positives de l'intelligence artificielle générative, il ne faut pas qu'elle loupe le coche en matière d'innovation comme de formation à ces nouveaux métiers. Les géants de la sont déjà dans les starting-blocks et, malgré l'existence de certaines start-up françaises prometteuses, notre pays et, plus largement, l'Europe font bien pâle figure face aux compagnies américaines et chinoises, qui investissent des milliards de dollars dans ces technologies. Ma première question, monsieur le ministre, porte donc sur les moyens que le Gouvernement compte mettre en oeuvre, pour, d'une part, soutenir l'innovation des entreprises françaises dans le domaine de l'intelligence artificielle, et, d'autre part, favoriser la formation à ces métiers d'avenir, ainsi que la reconversion pour les travailleurs dont l'emploi deviendrait obsolète. Abordons désormais certains aspects de l'intelligence artificielle générative qui sont autrement moins réjouissants que la hausse de la productivité et que la création de nouveaux emplois. Il apparaît en effet que des usages malveillants de ce type d'IA, ainsi que des erreurs du programme lui-même, peuvent avoir des conséquences dramatiques pour les libertés fondamentales, notamment le droit à la protection des données personnelles. Les expériences de ces dernières semaines, voire de ces dernières années, nous prouvent que ces dangers sont réels : qu'il s'agisse du non-respect du RGPD par ChatGPT, du jeune homme poussé au suicide par le chatbot Eliza en Belgique, des images devenues virales du Président de la République et du pape, créées par intelligence artificielle, des de personnalités publiques, du logiciel de recrutement d'Amazon qui discriminatoire envers les femmes, ou encore du scandale des allocations familiales aux Pays-Bas, où un algorithme d'auto-apprentissage ciblait les minorités et les accusait à tort de fraude, les exemples sont nombreux et se multiplient. découlent d'une non-conformité du logiciel avec la réglementation, d'erreurs faites par l'intelligence artificielle ou d'usages sciemment malveillants qu'en font ses utilisateurs, il est nécessaire de trouver des solutions et de légiférer pour éviter ces effets de bord, sans pour autant interdire les intelligences artificielles génératives. Il s'agirait en effet d'une grave erreur d'un point de vue économique, qui ferait une nouvelle fois perdre à la France du temps dans la course effrénée à l'innovation. Les entreprises développant des intelligences artificielles sont elles-mêmes en faveur de l'élaboration d'une réglementation, comme l'a récemment fait savoir OpenAI, car ce n'est qu'avec un cadre clair, assurant une assurant une sécurité juridique, que les potentialités économiques et sociétales de l'intelligence artificielle pourront pleinement se réaliser. Le RGPD apporte un premier échelon de réponse en matière de protection des données utilisées par les intelligences artificielles, mais il n'est pas suffisant pour éviter l'ensemble des potentielles externalités négatives et peut, parfois, se révéler contre-productif en matière d'innovation, notamment parce que ce n'est qu'en traitant certaines données personnelles que les entreprises pourront lutter contre les biais de certains systèmes d'intelligence artificielle. Des dérogations au RGPD devront donc être prévues, mais il faut qu'elles soient encadrées strictement pour nous prémunir de toute utilisation détournée de ces données sensibles, notamment à des fins commerciales. Ces dangers réels ou prévisibles des IA et cette inadaptation du RGPD ont conduit l'Union européenne à se saisir de la question des intelligences artificielles au sens large, par le biais d'une proposition de règlement.

Ce dernier est assurément un pas dans la bonne direction pour sécuriser les intelligences artificielles, mais mes corapporteurs et moi avons relevé certaines lacunes. Faute de temps, je ne m'arrêterai pas sur chacune d'entre elles, mais je souhaiterais, monsieur le ministre, connaître la position du Gouvernement sur nos propositions, ainsi que les points principaux que vous souhaitez soutenir au Conseil au sein de ce règlement. En outre, j'insiste sur l'absolue nécessité pour la France comme pour l'UE d'engager des discussions avec les pays tiers au sein des instances internationales de normalisation, pour les inviter à adopter des réglementations similaires. En effet, si nous sommes les seuls États à imposer des normes aussi ambitieuses, cela protégera certes les citoyens européens, mais cela pourrait nous désavantager d'un point de vue concurrentiel. Aussi, monsieur le ministre, pourriez-vous m'indiquer si des échanges ont déjà été entamés avec d'autres pays, notamment les États-Unis et la Chine, afin de promouvoir l'élaboration de législations similaires dans ces États ? La parole est à Mme Vanina

Au vu de l'accélération de ces technologies et des enjeux y afférents, nous avons jugé opportun de proposer de nouveau un débat sur ce thème. Je salue donc le choix collectif d'évoquer, ensemble, les défis de l'intelligence artificielle générative.

robotiser son outil logistique l'IA, ce qui permettra d'envisager la création d'une centaine d'emplois. Nous sommes à l'aube d'une vaste révolution de l'emploi et du rapport au travail. Cela vaut particulièrement pour les jeunes, qui sont plus que jamais en quête de sens dans leur vie professionnelle.

À ces inquiétudes, il nous faut répondre avec pédagogie, pour tirer profit des perspectives positives ouvertes par cette technologie. Il nous faut aussi répondre avec lucidité, pour anticiper les changements d'ampleur qui surviendront, notamment sur le marché du travail. Il nous faut enfin répondre avec fermeté, par un cadre réglementaire solide, pour garantir à nos concitoyens une intelligence artificielle fiable et sûre. L'Europe doit développer une approche éthique des données, avec une méthode et un cadre réglementaire propres.

La France est également pénalisée par la fuite de certains de ses cerveaux, alors même que leur formation a été assurée sur les deniers publics. Nous finançons, en partie, notre propre dépendance.

Les prochaines années s'annoncent décisives. Il n'est pas question de se laisser distancer davantage, sous peine de rater définitivement l'occasion de rester dans la course. Dès lors, monsieur le ministre, comment la France s'engage-t-elle pour ériger l'Europe en chef de file, tout en garantissant la sécurité et les droits des utilisateurs ? Que pensez-vous à cet égard des récentes positions de l'Italie ?

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, vous connaissez mon appétence pour l'intelligence artificielle. J'ai d'ailleurs moi aussi tenté de rédiger mon intervention avec ChatGPT, mais j'ai trouvé le résultat décevant. En revanche, je l'avais fait il y a quelques mois pour rédiger la question d'actualité que j'avais posée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse afin de l'alerter sur la suppression de la technologie en classe de sixième, alors même que cette matière est directement liée aux enjeux du numérique. En effet, la France a plus que jamais besoin d'une jeunesse ouverte aux sciences et aux technologies. En tant qu'enseignante, je suis impressionnée par les résultats obtenus par le recours à l'intelligence artificielle. Les perspectives semblent sans limites, dans des domaines aussi variés que l'agriculture, la logistique ou la santé.

je regarde avec intérêt la décision de l'Italie, qui vient de bloquer ChatGPT pour respecter la législation sur les données personnelles. L'interdiction n'est probablement pas la bonne solution, mais elle doit nous interroger sur les limites de cet outil. cet outil. Malgré la fascination que suscitent de telles innovations technologiques, nous devons garder les pieds sur terre et légiférer dans l'intérêt général. Il y a dix ans, nous nourrissions de grands espoirs vis-à-vis des assistants numériques comme Siri ou Alexa il y a encore quelques mois, nous parlions des cryptomonnaies avec des étoiles dans les yeux. Pourtant, ces innovations n'ont fait que créer de nouveaux besoins, sans apporter de solutions concrètes.

nous devons nous interroger sur les conséquences sociales d'un développement massif de l'intelligence artificielle. Dans une récente étude, Goldman Sachs estimait que 300 millions d'emplois seraient menacés par l'essor de l'intelligence artificielle. S'il ne sert à rien de crier au loup, nous ne pouvons ignorer cette alerte, d'autant qu'une partie des emplois qui sont créés par ces nouvelles technologies sont ingrats et mal payés.

Si l'intelligence artificielle ne remplace pas nos emplois, elle pourrait être à l'origine d'une nouvelle dégradation du travail. Enfin, l'intitulé de notre débat oublie un aspect fondamental, qu'il n'est plus acceptable d'ignorer au XX siècle

Derrière la chimère d'un numérique durable, dont les applications feraient disparaître par magie les risques environnementaux, il y a la réalité des chiffres. Ainsi, si les possibilités permises par l'intelligence artificielle nous font rêver, nous devons être pleinement conscients des impacts économiques, sociaux et environnementaux de cette technologie. L'intelligence artificielle est là, elle fait déjà partie de nos vies. Il n'est donc pas question de l'interdire ou de la réserver à une élite.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en 2018, le Grand Palais organisait une exposition intitulée « Artistes & Robots ». En 2019, c'était au tour du Barbican Centre, à Londres, de présenter au public une exposition interactive intitulée « ». À la curiosité et à l'enthousiasme suscités par l'émergence de ces nouvelles technologies, d'abord perçues comme récréatives et utiles en matière de productivité, ont succédé l'inquiétude, la méfiance et, surtout, les questionnements. Ne soyons pas dupes des intentions cachées de l'entrepreneur qui a orchestré la tribune tonitruante cosignée par plus de 1 000 experts du secteur de l'IA,

C'est d'ailleurs le sens de la décision de l'équivalent italien de la Cnil, qui a temporairement bloqué ChatGPT, pour deux motifs principaux. D'une part, aucun mécanisme de vérification de l'âge des mineurs n'est prévu, alors que le droit et la protection des mineurs en ligne sont un sujet politique majeur.

dont la fiabilité et la véracité peuvent être sujettes à caution, voire complètement fantaisistes. Ensuite, ces contenus pouvant être orientés, l'IA peut apporter des réponses comportant des biais importants, notamment sociaux, raciaux et de genre, ce qui peut avoir des conséquences dramatiques dans la formation des élèves et dans leurs Enfin, en l'état, l'usage d'IA génératives est contradictoire avec deux fondements essentiels de l'instruction, qui doit reposer sur des faits- et non de fausses informations -et favoriser l'acquisition d'aptitudes et de compétences

singulièrement à la définition de l'acte de création et à la protection du droit d'auteur. Sur ce point, je tiens à affirmer une position claire et sans ambiguïté : le cadre juridique, notamment européen, n'est ni adapté ni suffisant. Il est indispensable que, en cours de discussion au Parlement européen et percuté de plein fouet par l'émergence des IA génératives, comporte des dispositions qui protègent les artistes-auteurs. Au regard de la révolution que constituent ces IA, il n'est pas possible d'en rester à une simple possibilité pour les titulaires de droits qui ne souhaitent pas que leurs oeuvres alimentent ces machines. Le serait synonyme de déséquilibre et de renoncement à l'effectivité du droit d'auteur.

Ainsi, l'IA générative bouscule et interroge jusqu'à notre conception même de l'acte de création. Bien qu'elle en soit encore à ses prémices, il me semble que nous partageons l'intuition et la conviction qu'il nous faut impérativement l'encadrer, de sorte qu'elle soit porteuse du meilleur et non du pire. À nous de

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avec l'émergence de l'intelligence artificielle dans nos vies, le monde va vivre une quatrième révolution industrielle. Il la vit d'ailleurs déjà, des outils conversationnels ou de génération d'images particulièrement innovants et bluffants d'efficacité Nous aurions d'ailleurs tous pu demander à ChatGPT-4 de préparer ce discours- cela nous aurait fait gagner du temps. Au-delà du temps gagné, je pense que nous nous serions tous- ou presque -retrouvés avec le même discours, ce qui aurait rendu ce débat d'actualité fort ennuyeux.

Il y a donc de quoi avoir peur : que vont devenir les secteurs dont des milliers d'emplois pourront être remplacés efficacement par les intelligences artificielles ? Comment allons-nous apprendre, maintenant que l'intelligence artificielle est censée savoir faire à peu près tout ce qui demande de la réflexion ?

me fait penser à la phrase de la dirigeante de la- le patronat italien -Emma Marcegaglia : « Lorsqu'il y a une innovation, les Américains en font commerce, les Chinois la copient, et nous, Européens, nous en faisons un règlement. » En effet, le commissaire européen Thierry Breton a annoncé, avec une grande fierté, que, en moins de deux ans, l'Union européenne aura créé une réglementation pour encadrer les intelligences artificielles. Je vous avoue que j'aurais tout de même préféré qu'il annonce le lancement d'un grand projet de création d'un champion européen de Nous pouvons faire tous les règlements, toutes les lois, cette nouvelle révolution industrielle est lancée et elle ne pourra pas être arrêtée. Nous avons le choix de l'utiliser comme un merveilleux outil, notamment au service de la médecine et de l'éducation. Dans le monde du travail, les gains de productivité seront énormes.

Ma crainte est donc la suivante : n'avons-nous pas déjà pris trop de retard sur les entreprises américaines ? Aussi, monsieur le ministre, pouvez-vous nous rassurer sur le fait que la France sera au rendez-vous de cette quatrième révolution industrielle ? La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis quelques mois, les intelligences artificielles génératives influencent notre quotidien et monopolisent l'espace médiatique ChatGPT, Lensa ou Midjourney sont autant de logiciels d'IA engagés dans une course frénétique pour devenir la référence en la matière. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle générative ? Elle est un sous-domaine de l'intelligence artificielle, qui crée des contenus tels que des textes, des images, des vidéos, des programmes informatiques. C'est à l'IAG que l'on doit notamment les photos truquées du pape François en doudoune blanche ou de l'ancien président américain Donald Trump menotté, qui ont beaucoup circulé. Moins de deux mois après son lancement, en janvier 2023, ChatGPT, développé par l'entreprise californienne OpenAI, dépassait les 100 millions d'utilisateurs, ce qui en fait à ce jour l'application ayant connu la croissance la plus rapide.

L'intelligence artificielle est déjà en train de changer le monde du travail. Les machines sont capables d'apprendre et de s'adapter à des tâches qui étaient auparavant réservées aux humains. La question des conséquences sur l'emploi se pose, comme à chaque grande révolution technologique, ce qui déclenche appréhensions et crispations.

OpenAI a fait passer le concours du barreau américain à ChatGPT, qui a été brillamment reçu. Les experts de Goldman Sachs estiment ainsi que les IA génératives pourraient supprimer jusqu'à 300 millions d'emplois dans le monde. les grandes innovations ont souvent eu des conséquences sur les emplois. Le cabinet américain McKinsey souligne que le fossé risque de se creuser entre les travailleurs et entre les pays. Les principaux pays qui tireront parti de l'IA seront sans doute les États-Unis et la Chine. Toutefois, la France, le Royaume-Uni ou la Corée du Sud seraient relativement bien positionnés. D'un point de vue économique en général, l'IA générative peut avoir des impacts considérables. Selon les économistes de Goldman Sachs, l'adoption généralisée de l'IA pourrait accroître la productivité et augmenter le PIB mondial de 7 % par an. L'IAG, nous l'avons vu, peut être utilisée pour produire des contenus à grande échelle en un temps record ou pour créer des produits et des services personnalisés. Néanmoins, l'utilisation de l'IAG dans les affaires doit être éthique et responsable, afin de minimiser les impacts négatifs potentiels. Des propagées grâce à l'intelligence artificielle, des images truquées, de fausses révélations, peuvent avoir des répercussions très importantes sur les cours des Bourses mondiales et les faire chuter. D'un point de vue social ou sociétal, les effets de l'IA générative peuvent également se révéler positifs comme négatifs. Si celle-ci peut contribuer à la création de contenus artistiques et culturels innovants, elle peut aussi, par de faux contenus, semer la désinformation.

l'agence de police européenne Europol a averti que les criminels étaient prêts à tirer parti de l'intelligence artificielle. En somme, l'IAG peut avoir une incidence très importante sur la politique, en offrant de nouvelles aubaines.

russe Vladimir Poutine estimait dès 2017 que quiconque deviendrait le leader dans ce domaine deviendrait le dirigeant du monde. Aux États-Unis, Elon Musk, cofondateur d'OpenAI avec Sam Altman, l'inventeur de ChatGPT, a réclamé une pause de six mois dans la recherche sur l'IA, en évoquant « des risques majeurs pour l'humanité Le 4 avril dernier, le président Joe Biden a évoqué les risques liés à l'intelligence artificielle et a demandé au Congrès de fixer des « limites strictes » aux données personnelles collectées et d'interdire la publicité ciblée visant les enfants. En tant que pays leader en matière de technologie et de recherche, la France a un rôle important à jouer. Elle doit continuer de soutenir la recherche, tout en élaborant une réglementation adaptée, et investir dans la formation, tout en assurant la sécurité et la protection des droits des individus.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, j'ai suivi l'exemple de Monique de Marco et de Pierre-Antoine Levi en ne faisant pas appel à ChatGPT pour répondre à vos interventions- la preuve : papier, crayon

nous ne sommes donc ni technolâtres ni technophobes : nous considérons que la technologie doit être placée au service de l'homme. Certes, l'émergence très rapide de cette technologie suscite des questions

tous les moyens à nos concitoyens de se saisir de ces outils, afin qu'ils puissent en bénéficier. Nous devons nous assurer que l'adoption de ces technologies se fasse dans la justice sociale.

mérite d'être posée, la réponse apportée par les signataires de la récente pétition est mauvaise. À bien des égards, il nous faut accélérer, car la France dispose de tous les atouts pour maîtriser ces technologies d'intelligence artificielle générative.

des instituts interdisciplinaires d'intelligence artificielle (3IA) à Nice, à Toulouse, à Grenoble et à Paris, qui ont permis d'établir 190 chaires de recherche pour l'intelligence artificielle, de multiplier par deux le nombre de diplômés en intelligence artificielle

pour certains usages, le recours à l'intelligence artificielle sera proscrit. Pour d'autres, il sera encadré par des obligations de transparence et d'audit préalables à la mise sur le marché de ce type de solution. Pour d'autres encore, l'intelligence

la réglementation que nous construisons pour l'intelligence artificielle et celle que nous avons construite- et dont nous sommes très fiers -pour la protection des données personnelles. Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie du temps que vous avez consacré à ce débat.

est l'agenda dangereux, mais délibéré, d'examen de ce texte. Mes chers collègues, dans cette période de tensions sociales et politiques extrêmes, notre rôle de représentant de la Nation n'est pas de créer de la division. La violence que connaît notre pays et que nous condamnons est le symptôme d'une démocratie malade. Il n'est plus possible de voter des lois contre la majorité du pays ni de réprimer la contestation sociale par la force. Il nous faut donc appeler le pouvoir exécutif à l'apaisement, plutôt que de l'inviter à poursuivre sa dérive autoritaire et illibérale. Contrairement aux intentions des auteurs de cette proposition de résolution, ce n'est pas rendre service à nos forces de l'ordre, qui ne font que respecter les consignes de leur autorité. À l'opposé de cette démarche contre-productive, nous demandons au Gouvernement de faire des gestes d'apaisement pour protéger à la fois les forces de l'ordre et les manifestants. Nous lui demandons également de revoir de fond en comble la doctrine de maintien de l'ordre pour revenir à un usage proportionné de la force, afin de restaurer la confiance entre la police et la population. Pour toutes ces raisons, nous ne participerons pas au débat qui va s'ouvrir et nous ne prendrons pas part au vote.

de l'excuse, qui confine à une fascination pour le chaos, le désordre ou la violence. Ceux qui lancent des pierres cloutées sur les policiers, ceux qui brûlent

d'équivalence entre ce qui est illégitime et ce qui est illégal. Il ne saurait exister d'équivalence entre ce qui vise à protéger les citoyens, les biens ou les personnes

pour notre part choisi notre camp. Ce ne sera jamais celui du nihilisme, dans lequel une certaine ultragauche, voire une extrême gauche,

ce texte, ce ne sera clairement pas le cas. Quand bien même le Conseil constitutionnel s'intéresserait-il à cette proposition de résolution, je ne vois pas bien ce qu'il pourrait en dire.

Il ne leur serait pas venu à l'idée de me demander si je soutenais les forces de l'ordre, alors qu'ils savaient tous que j'étais de gauche. En outre, je vous rassure, ils ne m'ont même pas confondu avec un sympathisant de l'ultragauche Ils ne m'ont pas non plus demandé si je dénonçais les casseurs et, à aucun moment, je n'ai été accusé de terrorisme intellectuel. Notre assemblée a su montrer qu'elle savait voter des initiatives pour le bien commun, de résolution n'apporte rien au débat. Oui, la majorité des policiers et des gendarmes est exemplaire. Oui, le maintien de l'ordre est une matière difficile. Mais non, votre proposition de résolution ne prend pas en compte la réalité complexe des dernières semaines. Vous tentez de réduire la situation à un état de guerre de tous contre tous, bien manichéen. bien manichéen. Le Gouvernement doit bien sûr maintenir l'ordre. Là où nous percevons avant tout une immense colère sociale et une profonde inquiétude écologique relayées, pour l'essentiel, par des millions de manifestants pacifistes, vous ne retenez que les débordements, que nous condamnons également, de quelques dizaines d'abrutis dangereux armés de mauvaises intentions. En réalité, réalité, ce n'est pas la faute des manifestants si la pression ne redescend pas. Ce n'est pas la faute des manifestants si des journalistes se font parfois agresser par les forces de l'ordre. Ce n'est pas la faute des manifestants si l'on n'ose plus manifester en famille. Les responsabilités sont d'abord à chercher du côté du Gouvernement. À force de mépriser les corps intermédiaires, de nier l'utilité des syndicats ou de vouloir caricaturer les oppositions, l'exécutif a participé à la montée de la température sociale. Ce réchauffement politique, comme le réchauffement climatique, n'est pas inéluctable. Pour calmer les esprits, il faut entendre les avis contraires, prendre en considération les manifestants quand ils sont nombreux, éviter d'accroître la colère lors de passages au journal télévisé.

au rebut plusieurs centaines de milliers de signatures de citoyens, qui s'inquiètent de la manière dont le maintien de l'ordre est assuré en France. On n'est jamais gagnant quand on refuse le débat.

Selon un sondage Elabe du 29 mars dernier, 62 % des Français estiment que les violences policières sont marginales et que les dérapages sont le fait d'une minorité de policiers. À l'inverse, 37 % d'entre eux considèrent que ces violences ne sont pas marginales et sont représentatives d'un phénomène plus général au sein de la police. Je vous laisse disserter sur le verre à moitié plein ou à moitié vide.

de la tolérance et parfois de la bienveillance de certains responsables politiques à l'égard de ses auteurs », soulignez-vous. La violence « est aujourd'hui légitimée et encouragée par des élus qui tiennent des discours ambivalents ». En outre, « la violence physique est désormais précédée jusque dans nos institutions d'une violence verbale qui tente de justifier des comportements aussi illégaux qu'inadmissibles de ces points, vous avez raison s'il s'agit bien de dénoncer l'ultradroite et pas uniquement l'ultragauche, s'il s'agit de dénoncer les manifestations racistes à Callac

pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. » Nous appartenons à une famille politique qui a donné à la République de grands ministres de l'intérieur, Pierre Joxe figurant en tête. Nous croyons en une police issue des citoyens et au coeur de la société. Nous croyons en la police du préfet Grimaud, celle qui participe à la concorde républicaine, et nous savons pouvoir compter sur elle. Nous ne nous résignons pas à une police composée de fonctionnaires mal recrutés, insuffisamment formés et mal utilisés sur le terrain. vous avez choisi d'exprimer une gratitude inconditionnelle, souvent un peu pavlovienne, une gratitude d'ailleurs assez stérile pour les forces de l'ordre elles-mêmes. et Républicain, nous préférons exprimer notre soutien de principe, parce que nous ne sommes pas contre la police, et notre exigence de principe, parce que nous avons une haute idée du rôle républicain des forces de l'ordre. Cela nous permet d'exprimer notre inquiétude quand les circonstances l'exigent. C'est le cas en ce moment s'agissant du maintien de l'ordre.

Sans concertation, contre l'avis unanime des syndicats, contre une large majorité- qui n'a jamais fléchi -de l'opinion publique, sans entendre les mobilisations considérables et pacifiques pendant de longues semaines, le Président de la République tente d'imposer par la contrainte institutionnelle ce texte qui, pour ceux qui en subiront les effets, représente une violence considérable. L'obstination du Président de la République et de son gouvernement a durci le débat et a fait monter les tensions. Mesdames, messieurs de la majorité sénatoriale, nous vous appelons au sérieux et au respect. Nul à gauche de cet hémicycle ne souhaite la violence. Tant Chacun connaît la difficulté du métier de policier, de ces policiers détenteurs de missions de service public, qui doivent faire face à des situations créées par des choix politiques, dont ils ne sont nullement responsables. Vous le savez, c'est au soir du 49.3 que le climat a changé. La tension a atteint un sommet, la colère a explosé. C'est un fait, vous ne pouvez le nier. Des feux ont été allumés, des projectiles lancés, des membres des forces de l'ordre blessés et nous le regrettons, bien entendu. Nous avons toujours condamné- je l'ai toujours fait -l'action des groupes violents qui caricaturent et pourrissent le mouvement social. vrai ! Comment pouvez-vous fermer les yeux face à l'arrestation massive de centaines de jeunes « nassés », gardés à vue, dans des conditions juridiques contestables et contestées ? Combien de manifestants ont été blessés, parfois gravement ?

pour notre démocratie, une posture d'amalgame, de menaces voilées, de mise en cause de vos adversaires politiques sur un terrain inquiétant, celui de l'affrontement. Il n'existe pas de camps du bien et du mal, ni de l'ordre et du désordre. Vous ne représentez pas le camp du bien et de l'ordre, en ayant contribué largement à enfoncer notre pays dans la crise par votre vote sur ce projet de loi.

sommes-nous une menace à l'ordre public, quand nous alertons, aux côtés de nombreuses associations, dont la LDH, aujourd'hui menacée par le ministre de l'intérieur, sur des violences policières évidentes, étayées, constatées en France comme à l'étranger ? La République, mesdames, messieurs de la droite sénatoriale et de la majorité sénatoriale, ne se résume pas à l'ordre qui- c'est le moins que l'on puisse dire -n'a pas été son creuset. La République, c'est la démocratie et la justice sociale. Démocratie et justice sociale, c'est le projet que nous défendons aujourd'hui face à vous, que nous opposons à votre proposition de résolution profondément archaïque et réactionnaire, ... Tout en nuance ! ... raison pour laquelle nous ne prendrons pas part au vote.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, 1 143 : c'est le nombre de policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers blessés depuis le début des manifestations contre la réforme des retraites. À ce chiffre alarmant, derrière lequel se cachent tant de réalités humaines, s'ajoutent les 47 gendarmes pris en charge par les secours lors du dramatique épisode de Sainte-Soline, le 25 mars dernier. Depuis plusieurs années, les forces de sécurité de notre pays sont la cible d'un nombre inédit d'actes violents et brutaux. Dans le sillage des épisodes Notre-Dame-des-Landes et « gilets jaunes », ces agressions ont atteint un degré d'intensité rarement observé et particulièrement préoccupant. Ces violences sont souvent le fait d'individus instrumentalisant dangereusement le droit de manifester pour s'attaquer aux symboles et aux institutions de la République, quand il ne s'agit pas tout simplement de « casser du flic ces professionnels de l'affrontement violent nuisent à l'image de celles et ceux qui exercent très légitimement un droit fondamental de notre démocratie, celui de manifester. Pis, ils rendent impossible l'exercice serein de ce droit en s'attaquant volontairement à nos forces de l'ordre et aux services de secours. Nous n'aurons de cesse de défendre les femmes et les hommes qui protègent nos institutions et nos concitoyens. ce titre, je salue l'initiative conjointe des deux présidents des groupes de la majorité sénatoriale, Bruno Retailleau et Hervé Marseille, permettant l'examen aujourd'hui de la présente proposition de résolution. Celle-ci est un écho puissant à ce que de nombreux Français ressentent et constatent quotidiennement. En dépit de ce que veulent nous faire croire les professionnels de l'agitation et du désordre, les Français ne sont pas dupes. À l'occasion d'un récent sondage, 85 % des Français condamnaient les violences contre les forces de l'ordre. Personne ne nous fera croire que nous vivons dans un État policier. Personne ne nous fera croire non plus que nos forces de l'ordre sont des agents du chaos. Personne ne nous fera croire que nos policiers doivent « aller se faire soigner », pour reprendre les mots révoltants de M. Mélenchon. Mes chers collègues, il relève de notre responsabilité d'apporter un soutien clair et sans ambiguïté à ces femmes et ces hommes qui font la République au quotidien. Notre engagement à leurs côtés est total. Pour autant, il n'est pas aveugle. Dans le monde où nous vivons, policiers et gendarmes sont particulièrement exposés et soumis à une pression constante. Face aux provocations, aux insultes, aux crachats ou aux coups, des dérapages ont pu avoir lieu, inutile de le nier.

n'en demeurent pas moins isolés. De la même manière, il est normal que la justice ait été saisie après les affrontements de Sainte-Soline. Des personnes ont été blessées ; il est légitime qu'elles veuillent savoir comment on en est arrivé là. Si des incidents existent, ils ne reflètent en rien l'exemplarité et le sang-froid dont font preuve l'écrasante majorité de nos forces de l'ordre, alors qu'elles ont été particulièrement sollicitées, parfois plusieurs jours d'affilée, au cours des derniers mois. Quelques agitateurs de premier ordre aimeraient nous faire croire que, dans toute cette histoire, les casseurs sont les victimes et les policiers, les bourreaux ; que, sans gendarmes, il n'y aurait pas eu de dégradations à Sainte-Soline ; que, sans policiers, il n'y aurait pas eu d'incendie à la Encore une fois, les Français ne sont pas dupes. Ils savent que le maintien de l'ordre est un exercice très compliqué, qui impose parfois l'emploi de la force publique. Les appels à la dispersion ne suffisent pas toujours face aux jets de pavés, aux mortiers d'artifice, aux lancers de cocktails Molotov et de boules de pétanque. Bien sûr, l'utilisation des armes dont disposent les forces de l'ordre pour maintenir l'ordre doit être proportionnée et encadrée. Je pense notamment aux lanceurs de balles de défense (LBD) et aux grenades de désencerclement. Comme lors des manifestations des « gilets jaunes », nous avons vu resurgir des polémiques sur l'utilisation des LBD. Nous considérons que le problème n'est pas le LBD en lui-même : c'est l'usage qui peut malheureusement en être fait par des agents insuffisamment formés à son maniement. républicaines de sécurité (CRS) et gendarmes mobiles de cette arme intermédiaire sans proposer aucune solution de remplacement. De tels outils doivent être confiés à des professionnels du maintien de l'ordre, capables de les employer avec précision dans des situations complexes d'affrontement. Ces situations d'affrontement reflètent, dans tous les cas, l'échec d'un dialogue et l'achoppement d'une concertation. Pour autant, qui refuse le dialogue et la concertation dans notre pays ? Prenons l'exemple de Sainte-Soline. Tout se passe comme si les manifestants les plus radicaux incarnaient une forme de résistance à un pouvoir arbitraire, justifiant les violences dont ils se sont rendus coupables. Tout se passe comme s'il n'y avait pas eu d'études d'impact sur les mégabassines concluant à leur utilité dans l'adaptation au changement climatique et pour la souveraineté alimentaire de la France. Tout se passe comme si l'ensemble des parties intéressées n'avaient pas été entendues dans le cadre des comités de bassin et des commissions locales de l'eau, dont la représentativité n'est mise en doute par personne. Tout se passe comme si, à tous les niveaux de la gestion de l'eau, les responsables élus n'avaient pas tranché en faveur de l'aménagement des bassines, conformément au mandat leur ayant été confié. Tout se passe, enfin, comme si les convictions ou plutôt l'idéologie de certains devaient prévaloir, par la violence, sur des décisions de justice, sans que la police de la République puisse légitimement intervenir. Mes chers collègues, oui, les affrontements de Sainte-Soline incarnent une forme de résistance à l'arbitraire, mais la résistance de décisions démocratiques, confirmées par la justice et défendues par nos forces de l'ordre, à l'arbitraire d'une mouvance extrêmement violente,

je tiens également à adresser un hommage particulier à l'ensemble des agents qui participent aux secours et à la sécurité civile dans notre pays. Ils sont là pour protéger la vie de nos concitoyens : force est de constater que, pour cela, ils risquent chaque jour la leur.

Pourtant, sans ces sapeurs-pompiers et sans ces urgentistes, le bilan humain des manifestations serait autrement plus dramatique ! Par leur dévouement et leur sens du service, ils contribuent à apaiser la situation. C'est pourquoi, en responsabilité, en tant que défenseurs de l'ordre républicain, mes collègues du groupe Union Centriste et moi-même voterons en faveur de cette proposition de résolution, exprimant, par là même, notre profonde gratitude, notre reconnaissance et notre soutien aux policiers et gendarmes. La parole

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, après avoir oeuvré récemment, avec vous, pour la création de 200 nouvelles brigades de gendarmerie dans le pays, je tenais à prendre la parole pour exprimer ma gratitude et ma reconnaissance aux membres des forces de l'ordre déployées sur tout le territoire national, en particulier sur le territoire marseillais. Je tiens à saluer avec vous la mémoire d'Arnaud Blanc, gendarme du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN), tué le 25 mars dans une opération contre l'orpaillage illégal en Guyane. C'est dans cette même Amérique centrale et du Sud que l'extrême gauche dite française, ennemie de l'ordre et de l'autorité dans son propre pays, trouve ses meilleurs amis : les Chavez, Maduro, Castro, apôtres de l'effondrement économique, de la suppression des libertés fondamentales et de la répression policière sanglante. En effet, il faut dire les choses, si nous subissons un tel niveau de violence envers les forces de l'ordre, n'en déplaise aux falsificateurs et aux menteurs, c'est principalement l'oeuvre de la nouvelle union révolutionnaire des gauches, cette gauche des hémicycles qui légitime l'extrême gauche activiste et zadiste. À Paris, à Sainte-Soline, à Bordeaux, à Marseille, ils sont présents dans les rues et dans les facs, aux côtés de la racaille Antifa et autres Black Blocs. Nous avons vu cet ancien dealer, devenu député, cracher verbalement sur la police, tandis que des agents assuraient sa sécurité et protégeaient son domicile jour et nuit. Nous avons entendu M. Mélenchon en appeler à la « rééducation des policiers Il est temps de rappeler à Fidel-Hugo Mélenchon que « la République, c'est eux ! » Le Lider Maximo de l'islamo-gauchisme ferait mieux de se rééduquer lui-même et de rééduquer ses députés, qui hurlent aux prétendues violences policières, mais qui réintègrent l'un de leurs collègues qui frappe son épouse. M. Quatennens, on le sait, est pour que toute la France soit insoumise, sauf sa femme ... Quel argument ... Pour que la République et la France, surtout, ne sombrent pas dans le chaos auquel rêve et oeuvre la nébuleuse gauchiste, 6 700 policiers et 3 300 gendarmes ont été blessés en service en 2020. Le seul racisme systémique qui existe dans notre pays ... C'est le vôtre ! ... est le racisme anti-flics vociféré par une certaine gauche et l'extrême gauche. Cette haine des forces de l'ordre est largement partagée dans les cités de la diversité, où la police est perçue non seulement comme les représentants de l'ordre, mais aussi comme les représentants de la France que la racaille déteste plus que tout. Cette extrême gauche anarchiste anti-française embrigade les révoltés des causes sociales et du racisme anti-français pour en faire des soldats de la haine anti-flics. Notre pays, qui a vibré à la mort héroïque d'Arnaud Beltrame, est l'écrin précieux d'un processus de civilisation qui nous a transmis l'idéal chevaleresque. Ce sont ces figures d'abnégation qui fédèrent le pays et continuent d'écrire le récit national. Comme le 24 mars 2018, je salue ici tous ceux qui sont prêts à sacrifier leur vie pour protéger la nôtre. Cette proposition de résolution a le mérite d'identifier et de mettre face à face ceux qui se trouvent dans le camp de la Nation et ceux qui sont dans le camp de ses ennemis. Que chacun choisisse

pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.. je veux tenir ici une position sans équivoque : le groupe RDSE condamne sans détour tous les actes de violence commis notamment par des casseurs lors des manifestations qui ont eu lieu ces dernières semaines. Très largement, nous condamnons toutes les attaques portées à l'encontre des policiers, des gendarmes et parfois même des pompiers et de notre sécurité civile sur notre territoire. Tout le monde se souvient de l'hommage rendu aux forces de l'ordre pendant les manifestations contre le terrorisme en 2015. Nous étions déjà convaincus, avant ces drames, du courage et du dévouement de nos agents. Rien n'a changé depuis. Cependant, j'observe, chez certains de nos concitoyens, un sentiment de colère, de plus en plus tranché, un rejet de l'État et de la collectivité. J'aimerais toutefois redire à ceux qui doutent de l'intérêt de nos institutions qu'ils ne doivent pas oublier tous les services qu'elles nous rendent au quotidien. Policiers et gendarmes s'inscrivent dans un ensemble de services publics qui va des hôpitaux aux établissements scolaires, en passant par les réseaux routiers ou les services d'assurance chômage notamment.

Le rejet de toute autorité institutionnelle ne saurait être admis, en même temps qu'il doit nous interroger. Vivre en société, c'est aussi se soumettre à la contrainte sociale. Pour reprendre une formule du juriste bordelais Léon Duguit, « une société ne pourrait exister s'il n'y avait pas de discipline sociale, si une règle ne défendait pas certaines choses et n'ordonnait pas certaines autres aux individus qui la composent ». Je considère que la désobéissance civile n'est pas une option dans notre République et qu'elle est choquante quand elle est prônée par des élus, qui se devraient de la défendre. Elle est d'autant moins une option qu'elle est souvent sous-tendue par des idéologies douteuses, entre obscurantisme et complotisme. Nous n'y adhérons pas. Dans son exposé des motifs, la proposition de résolution indique qu'il est « inacceptable et dangereux de renvoyer dos à dos forces de l'ordre et casseurs ». Évidemment ! Toutefois, ne pas accepter la comparaison n'implique pas de renoncer à toute observation critique. Certaines images restent choquantes et peuvent mettre mal à l'aise. Il est possible d'être révolté face à l'incendie de la porte de la mairie de Bordeaux et de ne pas être absolument serein en voyant tourner en boucle des images de tirs de LBD et de jets de grenades. Oui, nous pouvons être reconnaissants du travail quotidien des agents de police et de gendarmerie, tout en nous inquiétant de la dérive d'une poignée d'entre eux lorsque nous entendons certains enregistrements. Cependant, s'inquiéter d'une augmentation, même marginale, des violences policières, c'est s'inquiéter, plus largement, de l'augmentation de la violence dans notre société. Il nous faut donc nous préoccuper de la santé mentale de nos agents, de leur état d'épuisement, des situations auxquelles ils sont confrontés quotidiennement. Il nous faut aussi veiller à ce que notre police soit irréprochable et que chaque dérive soit sanctionnée avec la plus grande fermeté. En notre qualité de parlementaires, nous devons les accompagner et les soutenir, par exemple en leur accordant les moyens nécessaires à l'exercice de leur métier dans des conditions décentes. En conclusion, mes chers collègues, le groupe RDSE veut réaffirmer avec force sa gratitude et sa reconnaissance aux membres des forces de l'ordre. Aussi, ses membres voteront pour cette proposition de résolution. La parole

j'aimerais à mon tour rappeler combien la place des forces de l'ordre est cruciale dans nos sociétés démocratiques, combien nous leur sommes redevables. Cette place a quelque chose à voir avec ce qui est au fondement de nos sociétés civilisées : le contrat social, lequel ne serait qu'un voeu pieux s'il n'y avait une force à même de le rendre exécutoire, de contraindre, au besoin par la coercition physique, les individus qui refusent de le respecter. C'est parce que nous savons qu'il existe une force capable d'imposer le respect des lois que nous pouvons jouir paisiblement de nos existences. La police apporte la force au droit. Elle arme l'ordre démocratique contre ceux qui voudraient s'y soustraire ou lui en substituer un autre, injuste et arbitraire. En somme, pour paraphraser Blaise Pascal, elle permet à ce qui est juste d'être fort. Sans police pour en assurer le respect, point de contrat social : le droit ne serait que de vaines taches d'encre sur d'insignifiantes pages de codes. c'est donc tout notre ordre social démocratique qui repose sur l'existence de cette force permettant d'éviter la « guerre de tous contre tous », comme l'a si bien décrit Thomas Hobbes. Que cela soit clair, manifester son soutien aux policiers et sa reconnaissance pour leur engagement ne revient pas à prendre parti contre la liberté de manifester. La rhétorique stérile qui voudrait dresser les manifestants contre les forces de l'ordre est inepte. Les unes sont là non pour entraver la liberté des autres, mais, au contraire, pour la garantir, notamment contre le noyautage des manifestations pacifiques par des perturbateurs qui y trouvent une couverture à leurs méfaits. C'est ce dernier risque qui, de nos jours, met le plus en péril à la fois la sécurité des manifestants et l'intégrité des forces de l'ordre. Avant l'irruption des Black Blocs dans les cortèges syndicaux, tous les observateurs relevaient le faible nombre d'incidents et saluaient le bon déroulement des rassemblements, la coopération des organisateurs. C'est donc aux agresseurs de policiers, aux incendiaires de poubelles, aux briseurs de vitrines, aux lanceurs de pavés qu'il faut jeter la pierre. Ils sont les seuls fautifs des effusions de violence que l'on a observées de Sainte-Soline à Paris. La réprobation à leur endroit doit être unanime. En effet, le droit de manifester n'est pas le droit à la chienlit. Qui pourrait en disconvenir ? Qui s'offusquera que la force doive rester à la loi ?

la non-violence. La seule liberté alors reconnue est celle de « s'assembler paisiblement et sans armes, en satisfaisant aux lois de police dans le respect de « la liberté d'autrui et de la sécurité publique ». Cette conciliation entre liberté et ordre public est un invariant dans notre tradition juridique. Elle structure la façon dont notre droit conçoit l'étendue et les limites de la liberté de manifester. Devrions-nous considérer avec mansuétude les violences des Black Blocs et pousser des cris d'orfraie lorsque la police intervient pour y mettre fin ? Quel triste enchantement a conduit certains esprits à cette inversion des coupables et des victimes, des fauteurs de troubles et des gardiens de la paix civile ? Qu'est-il reproché à la police ? De riposter lorsque l'on s'en prend à elle ? De se défendre lorsqu'un millier de ses agents sont blessés, plus ou moins gravement, par des assauts pénalement et moralement inacceptables ? Lui en veut-on de ne pas abandonner nos rues à une poignée de casseurs ? De s'interposer lorsque des commerces sont saccagés ? D'escorter des pompiers venant éteindre des incendies ? Ce que ses contempteurs reprochent à la police, c'est bel et bien de ne pas désarmer face à une violence qu'ils cautionnent peut-être dans le secret de leurs coeurs. Ils blâment la police de faire ce pour quoi elle a été instituée : préserver l'ordre républicain établi par les lois que notre société s'est prescrites au travers de ses institutions démocratiques. Ce faisant, ils répudient le contrat social qui nous lie. C'est pourquoi nous devons, nous autres sénateurs, témoigner notre gratitude envers les défenseurs des droits que sont les policiers et leur redire notre confiance quand traîner la police dans la boue, la couvrir d'accusations infamantes est devenu le fonds de commerce médiatique d'une partie de la classe politique. Non, nous n'accepterons pas que le bruit et la fureur soient des codicilles au contrat social. Non, les CRS n'ont pas vocation à devenir de la chair à Black Blocs. Non, nous ne laisserons pas la police être livrée à quelque vindicte que ce soit dans l'opinion publique. Sans bouclier, nous sommes faibles. Toute démocratie le sait

CRCE. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous avons assisté, ces dernières semaines, à un véritable déchaînement de violence dans notre pays. Des mairies ont été incendiées. De très nombreux parlementaires ont été la cible d'attaques, y compris dans leur domicile. On ne compte plus les devantures de magasins et les véhicules incendiés et détruits. Voilà l'image que nous livrons au monde. Chaque jour de manifestations, les forces de l'ordre affrontent des individus armés, décidés à casser, à incendier, voire à tuer. Ce sont des cocktails Molotov, des boules de pétanque et des battes de base-ball qui ont été employés contre nos policiers et nos gendarmes le 26 mars dernier à Sainte-Soline- tout cela bien évidemment pour une manifestation non violente ... Force est de constater que l'ultragauche attaque aujourd'hui délibérément notre République et notre démocratie. La France doit cesser d'être la terre de jeu européenne de ces factions extrémistes. Les mouvements d'ultragauche doivent être démantelés. Il faut lutter contre la complaisance intellectuelle et politico-médiatique envers ces groupuscules. La réponse pénale en cas d'agression contre un dépositaire de l'autorité publique doit absolument être renforcée dans notre pays, afin d'être enfin dissuasive. Ceux-là mêmes qui avaient promis de transformer l'Assemblée nationale en zone à défendre (ZAD) ont empêché le débat démocratique par une guérilla indigne du Parlement et sont aujourd'hui dans la rue aux côtés des casseurs. Les Français ont des opinions diverses. Il est un point sur lequel ils sont néanmoins accordés, c'est que la démocratie doit nous gouverner. « Ce qui préserve de l'arbitraire, c'est l'observance des formes », disait Benjamin Constant. En tant que représentants de la Nation, il est de notre devoir de réaffirmer que la violence n'est pas un moyen d'expression légitime dans notre démocratie et dans notre République. Nous avons et nous aurons des désaccords : c'est normal. Les gouvernements feront toujours face à une opposition : c'est naturel et c'est là le principe de la démocratie. Il importe cependant que cette opposition s'exprime par la voie démocratique. Alors que notre pays connaît des accès de violence, je veux rendre hommage, au nom du groupe Les Indépendants - République et Territoires, aux hommes et aux femmes qui dédient leur vie à la protection de nos concitoyens et de nos institutions. Ce sont eux qui protègent la France contre la délinquance et le terrorisme, eux qui sécuriseront les grands événements que notre pays s'apprête à accueillir, eux encore qui doivent faire face aujourd'hui à une violence encouragée par quelques irresponsables politiques. Prises pour cible par des révolutionnaires de salon, les forces de l'ordre le sont ensuite dans la rue. Depuis le début des manifestations, on compte plusieurs centaines de blessés- il y en a eu 154 pour la seule journée de jeudi dernier. dernier. Malgré l'intensité des tensions, malgré le risque qu'ils encourent, nos policiers et nos gendarmes continuent d'exercer leur métier avec un grand professionnalisme. Avec courage et sang-froid, ils font face à des individus qui cherchent en permanence à provoquer l'embrasement. À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation, je veux, au nom de mon groupe, leur dire qu'ils peuvent compter sur notre soutien. Nous exprimons, aujourd'hui encore, notre reconnaissance aux gardiens de l'ordre républicain. Contrairement aux manifestants, la police et la gendarmerie ne sont les défenseurs d'aucune idéologie. Ils sont au service de tous les Français et de nos institutions républicaines.

Monsieur le président, la proposition de résolution que nous examinons aujourd'hui est certainement révélatrice d'un climat social et politique que notre pays connaît depuis une vingtaine d'années. En effet, s'il y a bien un constat que nous partageons, c'est que les contestations auxquelles notre pays est confronté sont de plus en plus violentes. Ces phénomènes de violences ne touchent pas que la France. Rappelez-vous ces scènes de guérillas et d'émeutes lors du G20 de Hambourg en 2017, avec trois jours de déferlement de violence et de haine. le G8 de Rostock, en 2007, où l'on a compté plus d'un millier de blessés, ou encore le G20 de Londres. L'apparition des zones à défendre, les fameuses ZAD- en réalité, de véritables zones de non-droit -est également devenue un phénomène récurrent. chez nos voisins, il y a eu, au mois de janvier 2023, à Lützerath, en Allemagne, de violents affrontements, au cours desquels les policiers ont essuyé des tirs d'engins pyrotechniques et des jets de projectiles, faisant plus de 70 blessés.

Cette mouvance internationaliste touche également la France. Cette nouvelle génération d'activistes d'ultragauche, ou d'ultradroite, se structure au printemps 2006, lors de la mobilisation contre le méprisent les mobilisations institutionnelles. Ils méprisent les manifestations encadrées. Ils encouragent l'insurrection et profitent des contestations pour semer le chaos. Plusieurs lieux de forte contestation sont devenus tristement célèbres

Depuis, nous le voyons bien, du mouvement des « gilets jaunes » jusqu'à la mobilisation contre la réforme des retraites, l'ultragauche et l'ultradroite infiltrent toutes les revendications pour les radicaliser. Nous pouvons observer que ces contestations entretiennent des liens entre elles, mais également avec des mouvances étrangères. Ainsi, à Sainte-Soline, les forces de l'ordre ont également été confrontées à des éléments radicaux venant d'Italie, d'Allemagne ou encore de Belgique. D'ailleurs, selon la préfète des Deux-Sèvres, « tout porte à croire que les activistes violents visaient davantage les forces de l'ordre pour elles-mêmes et, à travers elles, les institutions républicaines Personne, et surtout pas les organisateurs, ne pouvait alors ignorer la violence qui se déchaînerait lors du rassemblement qu'ils avaient préparé. Le directeur général de la gendarmerie nationale a indiqué que les éléments radicaux avaient pour objectif de « mettre en échec la capacité des gendarmes à maintenir l'ordre public et à assurer la protection des institutions ». Je le dis avec gravité, mes chers collègues, on ne peut que regretter la duplicité de certains membres de notre Parlement. Ces élus portent une lourde responsabilité, par leur attitude, leurs propos et leur silence. Des noms ! En participant à ces manifestations interdites, en ne condamnant pas clairement les violences à l'encontre de nos forces de l'ordre, ces élus jouent un jeu dangereux.

Si le groupe RDPI salue et votera pour cette proposition de résolution exprimant la gratitude et la reconnaissance du Sénat aux forces de l'ordre, je tiens à rappeler que le renforcement des moyens, l'amélioration des conditions de travail et la revalorisation des carrières sont la meilleure preuve de gratitude et de reconnaissance que l'État puisse fournir aux forces de sécurité intérieure. Le premier quinquennat du Président Macron a été marqué par un renforcement considérable des moyens alloués au ministère de l'intérieur, avec, je le rappelle, 10 milliards d'euros de budget supplémentaires, 10 000 policiers et gendarmes recrutés, le renouvellement de la moitié du parc automobile, le paiement de plusieurs millions d'heures supplémentaires cumulées non rétribuées durant plusieurs années. 2023 est la première année de mise en oeuvre des mesures prévues par la loi du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, la fameuse Lopmi. Ce texte prévoit un renforcement et un effort budgétaire inédit, de 15 milliards d'euros, entre 2023 et 2027, ce qui permettra notamment le doublement de la présence des forces de l'ordre sur le terrain d'ici à 2030. À cette fin, le ministère de l'intérieur bénéficiera de 8 500 créations d'emploi d'ici à 2027- en plus des 10 000 emplois que nous avons créés lors du précédent quinquennat. Rien que cette année, les effectifs des forces de l'ordre seront augmentés de 2 857 emplois à temps plein. Ces nouveaux gendarmes et policiers

Plusieurs mesures sont par ailleurs prévues pour renforcer l'accompagnement social des personnels et de leurs familles : amélioration des aides aux blessés et de l'aide à la reconstruction par le sport, densification du réseau de psychologues cliniciens

dans cet hémicycle que nous apportons un soutien concret, plein et entier aux forces de l'ordre. Au nom du groupe RDPI, nous exprimerons clairement notre pleine reconnaissance et notre gratitude aux forces de l'ordre en votant cette proposition de résolution.

madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, jusqu'à la mi-mars, à l'appel de l'intersyndicale, les manifestations contre la réforme des retraites se déroulaient un peu partout sur le territoire de manière organisée et pacifique. Manifestants, Gouvernement ou médias se félicitaient du bon déroulement de cet exercice d'un droit démocratique. Pourtant, le 16 mars dernier, la décision de la Première ministre de recourir au 49.3 a été le point de départ de violences urbaines, qui ont ensuite émaillé toutes les manifestations, notamment celle du 23 mars ou encore celle du 5 avril dernier. Nous avons assisté, le 25 mars dernier, dans un autre contexte, à un déchaînement de violence à Sainte-Soline, alors même que la manifestation était interdite sur le site des retenues d'eau. Le bilan de ces mois d'affrontements est lourd : près de 2 000 interpellations, plusieurs centaines d'atteinte à des institutions de la République, plus de 1 300 policiers, gendarmes ou pompiers blessés, 2 500 incendies sur la voie publique, dont certains menaçant certains immeubles et leurs habitants. Ainsi, un drame a été évité de peu à Paris, où des personnes, notamment des enfants, ont dû être évacuées par nos forces de sécurité. Face à ce chaos, elles ont fait preuve d'un grand sang-froid pour assurer malgré tout leur mission de protection des biens et des personnes. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons leur rendre hommage et leur apporter tout notre soutien aujourd'hui. Il s'est pourtant trouvé plusieurs élus, membres de diverses associations prétendument humanitaires, pour se livrer à une mise en cause indécente des policiers et des gendarmes, les accusant de brutalité et de violence à l'égard des manifestants. Nous avons assisté ici même à un renversement des valeurs, les agresseurs devenant les agressés. Nos forces de l'ordre ont dû contenir les assauts répétés de certains indignés professionnels, qui ont été qualifiés de « simples promeneurs Depuis quand les personnes qui souhaitent manifester ou protester doivent-elles s'équiper de cocktails Molotov, de boules de pétanque, de marteaux, de battes de base-ball, de manches de pioche ou de pavés ? À Sainte-Soline, cet arsenal qualifié de « festif » était complété par des bombonnes de gaz, des aérosols, des bidons d'essence ou encore des mortiers d'artifices. Certains étaient manifestement venus dans l'intention de « taper du flic », encouragés par des slogans stupides comme « la police tue ». Les fourgons en feu de la gendarmerie ne laissaient pas de place au doute quant à leur détermination à en découdre.

Leur objectif : attaquer et détruire la société capitaliste et ses institutions républicaines, jugées intrinsèquement bourgeoises. Nos services de renseignement ont confirmé une stratégie d'infiltration des mouvements sociaux, en oeuvre par l'ultragauche dès la mi-mars, afin de faire basculer des manifestations pacifiques en soirées d'émeute contre tout symbole de l'État et, en premier lieu, contre ces représentants de l'ordre républicain que sont les policiers et les gendarmes. Cette violence n'a rien de symbolique. Les vitrines des banques, des assurances, des McDonald's ou encore des grandes enseignes de commerce en ont elles aussi fait les frais. Pour cette mouvance, le recours à la violence doit susciter un processus dit insurrectionnel,

République. Nous avons constaté l'impossibilité pour cette mouvance, qui se dit pourtant démocrate, de condamner clairement les violences exercées contre nos forces de l'ordre. Nous l'avons vu à Sainte-Soline : elle invoque le droit de manifester,

Bruno Retailleau a déposé une proposition de loi qui, au terme de son parcours législatif, a donné naissance à la loi du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre lors des manifestations. Malheureusement, une décision du Conseil constitutionnel est venue remettre en cause l'application de ce texte,

notre reconnaissance aux forces de l'ordre. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, depuis plusieurs années l'activité des forces de l'ordre s'est considérablement accrue sur le territoire métropolitain.

Cette agitation permanente met les forces de l'ordre en tension, éreinte les personnels et complique leur vie familiale. On ne compte plus leurs heures supplémentaires ni les blessures, parfois graves, qu'elles subissent pour assurer la sécurité des Français et faire appliquer les lois.

Cette violence peut être encore amplifiée par des flux migratoires incontrôlés qui créent des situations explosives, comme c'est le cas à Mayotte. En Guyane, l'immigration illégale venue du Brésil ou du Surinam accentue la prédation sur les ressources : pêche illégale, coupe de bois, orpaillage, pollution des sols et des cours d'eau, etc. Nos forces y travaillent dans des conditions difficiles et dangereuses. Un gendarme d'élite y a d'ailleurs perdu la vie il y a quelques jours. Le trafic de drogue, particulièrement de cocaïne, vers la métropole mobilise aussi policiers, gendarmes et douaniers. Aujourd'hui, nous exprimons notre reconnaissance aux forces de l'ordre. C'est d'autant plus nécessaire qu'elles font face à des individus de plus en plus radicalisés et désinhibés,

que cette violence est globale et ne vise pas que la police ou la gendarmerie. Sont aussi ciblés de nombreux agents du service public- des médecins, des pompiers, des enseignants, des élus nationaux ou locaux.

Je pense tout autant au désespoir d'une partie de notre jeunesse, entre perte de repères et écoanxiété, et à celui des territoires périphériques en voie de paupérisation, dont le mouvement des « gilets jaunes » était en fait l'expression.

de la liberté. Il faudra s'attaquer rapidement à ces problèmes pour éviter que la violence ne se déchaîne systématiquement sur les forces de l'ordre et n'aboutisse à des tragédies que- je le crois -personne ici ne souhaite. La parole

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, avant tout, permettez-moi d'avoir une pensée émue pour le gendarme Yannick Pierre et l'adjudant de réserve Patrick Hervé, décédés hier au cours d'une opération de lutte contre la délinquance routière,

l'ordre s'engagent pour la France et les Français : à Paris, pour garantir la liberté de manifester ; à Sainte-Soline, pour lutter contre ceux qui tentent de mettre à genoux notre République ; à Nouméa, à 22 000 kilomètres de la métropole, pour honorer la parole de la France dans les outre-mer. Que les femmes et les hommes qui constituent les forces de sécurité intérieure soient assurés de l'entier soutien et de la totale reconnaissance du ministère de l'intérieur et des outre-mer. Ces forces sont les seules garantes de l'ordre public, de l'ordre républicain, du seul ordre qui vaille. Leur rôle est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui précise en son article XII : « La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous. » Cette force, ce sont les femmes et les hommes qui s'engagent au quotidien pour la sécurité des Français. des Français. C'est la force qui garantit le droit à la liberté contre ceux qui veulent saper le fonctionnement de nos institutions et de notre démocratie ; la force qui garantit le droit à la propriété contre ceux qui brûlent les voitures, les immeubles et les portes de mairie la force qui garantit le droit à la sûreté et l'ordre républicain contre ceux qui pratiquent la guérilla urbaine et s'en prennent aux outils de travail de nos agriculteurs, à nos commerces, bref aux honnêtes travailleurs.

aux Antilles, pour lutter contre l'insécurité et le trafic de drogue, qui gangrènent le territoire, ou en Guyane, pour combattre les cartels et les orpailleurs. J'ai d'ailleurs une pensée émue pour le major Arnaud Blanc, mort dans l'exercice de ses fonctions, dans cette lutte de chaque instant contre ceux qui pillent et détruisent sans vergogne le territoire guyanais. Nos forces de l'ordre interviennent également à Mayotte pour freiner l'immigration comorienne, qui place nos concitoyens mahorais dans une situation insoutenable. Dans le Pacifique enfin, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna ou en Nouvelle-Calédonie, elles sont engagées sur un large spectre de missions et concourent, entre autres, à la préservation du fragile écosystème qui fait la richesse de nos îles océaniennes. Pourtant, ces dernières semaines, ceux-là mêmes qui garantissent l'État de droit et la sécurité de tous les Français ont été la cible d'attaques inacceptables. Cocktails Molotov, pavés, insultes, appels à la haine depuis le 19 janvier dernier, première journée de mobilisation contre la réforme des retraites, nous assistons à une montée en puissance de la violence à l'encontre de nos forces de l'ordre. Plus de 1 800 policiers et gendarmes ont été blessés depuis cette date, dont 1 381 au cours des quatre dernières semaines.

Ne nous y trompons pas : cette violence cherche à fracturer la société en s'attaquant aux institutions de la République, en discréditant les forces et l'ordre et en contestant la légitimité parlementaire. Notre Il ne saurait être à géométrie variable. Le devoir de nos forces de l'ordre est avant tout de permettre l'exercice de la liberté de s'exprimer lors de manifestations déclarées et autorisées.

étant formulé, nous avons toutes et tous constaté l'extrémisme de groupuscules dont les membres sont responsables de grandes violences. Je pense notamment à un certain groupement, Les Soulèvements de la Terre, dont les membres ont envahi des entreprises, commis des exactions graves contre les forces de l'ordre, détruit nombre de biens et lancé plusieurs appels à l'insurrection. Face à ces organisations factieuses, la main du Gouvernement ne tremble pas. Nous avons pris les mesures qui s'imposent pour maintenir l'ordre dans notre pays. C'est pourquoi Gérald Darmanin a engagé la dissolution de ce groupement. Je puis vous assurer de la pleine mobilisation des services de renseignement pour anticiper et détecter la formation et les actions de groupuscules, d'ultragauche comme d'ultradroite, ... Il est bon de le

Nous avons pris toutes les mesures qui s'imposent pour appréhender ces fauteurs de troubles. Un vaste travail a été mené pour rénover la doctrine du maintien de l'ordre. Le nouveau schéma national, qui tient compte des évolutions de la sociologie revendicative et met davantage l'accent sur la relation avec les manifestants, a d'ores et déjà des effets encourageants. Le déroulement des dernières manifestations témoigne de la juste adaptation de ces nouveaux dispositifs, notamment en milieu urbain. Certes, il y a eu des dégradations, mais nous ne déplorons aucun incident majeur.

des réserves opérationnelles de la gendarmerie et de la police vont, par ailleurs, être portés respectivement à 50 000 et 30 000 personnes. Les agents vont aussi bénéficier de matériels et de tenues modernisés et le parc automobile des forces de l'ordre va être renouvelé au rythme annuel de 10 %. En outre, en vue des jeux Olympiques et Paralympiques que la France accueillera en 2024, onze nouvelles unités de forces mobiles (UFM) seront déployées cette année et l'année prochaine sur l'ensemble du territoire. Parallèlement, sept UFM seront rendues disponibles par la reprise des sites par les préfectures de police. Soyez assurés de la mobilisation pleine et entière du ministère dans la préparation de cet événement majeur pour notre pays. Il y va de l'honneur de la France : nous devons garantir aux forces de l'ordre les moyens d'exercer leurs missions avec dignité et sérénité, au service de la République et de la démocratie. La confiance des Françaises et des Français envers les forces de l'ordre et le soutien que nous leur apportons n'entame en rien l'exigence de déontologie et de respect du droit que nous leur assignons et à laquelle ils s'astreignent. Le corollaire de cette mission au service de la République, c'est l'exemplarité : chaque fois qu'un policier dérape- cela peut arriver -, c'est la relation des citoyens aux forces de l'ordre, au ministère de l'intérieur et même à la République qui se dégrade. S'il arrive que des policiers et des gendarmes sortent du cadre fixé par la loi, si l'équilibre entre nécessité et proportionnalité n'est pas respecté, des enquêtes sont menées et les responsables sont évidemment sanctionnés.

Tenir un autre discours reviendrait à jeter l'opprobre sur ces ouvriers de la sécurité que sont nos policiers et nos gendarmes. Gérald Darmanin et moi-même, nous mesurons ce que les gendarmes et policiers accomplissent au quotidien, ce que cela représente pour eux d'engagement, d'abnégation, de courage et de sacrifices. J'ai d'ailleurs une pensée particulière pour leurs familles et leurs proches, qui, eux aussi, portent le poids de cet engagement. Ces femmes et ces hommes méritent toute notre estime, toute notre reconnaissance. Les Françaises et les Français savent bien ce qu'ils leur doivent. Ils savent le rôle essentiel que jouent les forces de l'ordre pour leur permettre de mener une vie paisible : nous en sommes convaincus.

Le scrutin est clos.

la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a émis, lors de sa réunion de ce jour, un avis défavorable- 12 voix pour, 24 voix contre -à la nomination de M. Boris Ravignon à la présidence du conseil d'administration de l'Agence en application des mêmes dispositions, la commission des affaires sociales a émis un avis favorable- 21 voix pour, aucune voix contre -à la nomination de M. Lionel Collet à la présidence de la Haute Autorité de santé et la commission des affaires étrangères un avis favorable- 26 voix pour, aucune voix contre -à la nomination de M. Gilles Andréani à la présidence de la Commission du secret de la défense nationale. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, 471 jours nous séparent de l'ouverture des jeux Olympiques, le long de la Seine. Cette rencontre sportive hors norme se doit d'être une belle fête et chacun doit pouvoir profiter du spectacle en toute sécurité.

ce sens, le Sénat a multiplié les garde-fous, les contrôles et les garanties. Notre assemblée ne signe ni un chèque en blanc ni un chèque en gris aux autorités publiques. Nous cherchons à leur offrir les moyens et les capacités d'organisation nécessaires pour éviter d'autres épisodes regrettables.

Ainsi, le Sénat s'est attaché à garantir l'opérationnalité d'outils comme la vidéoprotection intelligente, les scanners biométriques, les tests génétiques pour la lutte antidopage ou encore le criblage. Leur caractère constitutionnel a été un souci permanent. Le Sénat a particulièrement veillé à la préservation de l'équilibre actuel entre le maintien de l'ordre public et la protection des libertés. C'est le sens du renforcement des garanties que j'évoquais Le développement de la vidéoprotection, qui a concentré notre attention, confirme la qualité du compromis trouvé entre les assemblées. La protection des droits des personnes a été le ciment de notre discussion.

Dans la foulée, nous sommes parvenus à un accord sur le terme de l'expérimentation, la durée de conservation des données d'apprentissage et la priorité accordée aux entreprises répondant aux exigences de protection en matière de cybersécurité. cybersécurité. Après avoir constaté le renforcement du dispositif des tests génétiques, lesquels sont essentiels pour respecter nos engagements internationaux, nous avons concédé un assouplissement des conditions de contrôle des sportifs entre cinq et six heures du matin.

La billetterie électronique est un autre acquis dont le Sénat peut revendiquer la paternité. C'est aussi l'une des leçons tirées des événements du Stade de France. Par ailleurs, l'articulation entre la mesure administrative d'interdiction de stade et la peine complémentaire, introduite par l'Assemblée nationale, a été conservée. Elle a paru cohérente avec la sécurité des enceintes sportives. Pour ce qui concerne l'autorisation préfectorale de dérogation des commerces au repos dominical, la procédure de l'Assemblée nationale, en deux étapes, a été retenue pour éviter les risques de contentieux. Toutefois, un assouplissement des modalités d'extension a été prévu. Enfin, les mobilités ont été un sujet de discussion. Je pense en particulier aux questions d'accessibilité pour les personnes utilisatrices de fauteuil roulant. Le seuil des dix autorisations de stationnement exploitées dans la zone de compétence du préfet de police de Paris a été supprimé. (CMP) a maintenu la possibilité d'imposer un signe distinctif pour reconnaître facilement les taxis accessibles aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant. pour toutes ces raisons, je vous invite à adopter ce texte, fruit d'un compromis parlementaire de bon sens, afin de résoudre des problèmes concrets d'organisation tout en faisant place à l'innovation dans le respect des libertés.

c'est un réel plaisir pour moi de revenir devant le Sénat au lendemain du vote par l'Assemblée nationale des conclusions de cette commission mixte paritaire, dont je tiens à souligner le succès. Il démontre

à nous fixer des objectifs communs et à trouver les bons équilibres sur certaines problématiques sensibles. Je pense aux mesures de lutte contre les violences et les incivilités dans nos stades. Je pense également à la conciliation que nous avons recherchée, en matière de sécurité,

de nos engagements internationaux. Le texte issu de nos travaux satisfait ainsi aux impératifs que nous avions conjointement établis. Il reste centré sur l'essentiel ; à preuve, il compte moins de trente articles. Il contient toutes les mesures indispensables au bon déroulement des Jeux. Il est intégralement orienté vers la phase opérationnelle opérationnelle de notre préparation collective, tout en assurant le plein respect des droits et libertés de nos concitoyens. Ce texte couvrira ainsi l'ensemble de nos objectifs sans renoncer à nos principes une polyclinique et des professionnels de santé, mobilisés au service des athlètes et des délégations, sans monopoliser les moyens de notre système de santé ni diminuer notre offre de soins ; une nouvelle dynamique donnée à la formation aux gestes qui sauvent, pour développer chez nos concitoyens le sens de l'engagement et du premier secours ; une lutte contre le dopage qui demeurera aux meilleurs standards internationaux. Le processus parlementaire a également permis de doter nos policiers et gendarmes d'outils plus modernes pour assurer de meilleures conditions de sécurité et de coordination opérationnelle, lors de nos grands événements sportifs. Le renforcement du cadre juridique relatif au traitement des images

cadre de la navette. Enfin, notre texte va permettre de faire vivre ces Jeux dans l'ensemble de nos territoires, en métropole comme en outre-mer, avec des animations festives, tout au long du relais de la flamme et une activité commerciale le dimanche, du 15 juin au 30 septembre 2024, à proximité de nos sites de compétition. Plus globalement, ce texte fait vivre les exigences que nous promouvons dans notre modèle des grands événements sportifs : l'impératif d'accessibilité des sites et des transports au service d'un regard nouveau porté sur le handicap ; des mesures fortes au service de notre responsabilité environnementale, notamment en termes de mobilité durable

et d'une recherche constante d'efficacité. Cela démontre, comme je le disais hier à l'Assemblée nationale, que lorsqu'il s'agit de faire réussir la France en organisant le plus impeccablement possible le premier événement sportif planétaire, il n'est de clivages partisans qui ne sauraient être surmontés. Dès que cette loi sera- je l'espère -adoptée et promulguée, j'aurai à coeur, avec mes collègues, en particulier Gérald Darmanin, Clément Beaune et François Braun, d'assurer sa mise en oeuvre dans les plus brefs délais. Nous avons amorcé ce travail et le poursuivrons sans relâche

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons une dernière fois cette loi improprement appelée « olympique », puisqu'il n'y est question ni de sport ni de transmission des valeurs olympiques. Nous ne pouvons que continuer de déplorer le caractère strictement sécuritaire Le sport aurait dû nous inspirer la liberté ; nous en sommes aux antipodes. Sous prétexte d'assurer la sécurité des Jeux, ce qui est bien nécessaire, les dispositions attentatoires aux libertés et aux droits fondamentaux du texte proposé par la commission mixte paritaire vont s'inscrire dans la durée, alors même que rien n'a encore été sérieusement programmé pour l'héritage sportif du pays. Le projet de loi est bien loin d'honorer les principes universels et fédérateurs des jeux Olympiques. À titre d'exemple,

Le sport fait pourtant appel à des valeurs universelles de respect, de partage, de refus des discriminations, d'égalité et de fraternité. Comme il est dommage de les mettre en marge de l'esprit qui gouverne les jeux Olympiques de Paris L'inscription dans la loi d'une telle campagne de prévention aurait eu tout son sens au nom de l'esprit olympique et nous ne nous satisfaisons pas de l'argument selon lequel ce souhait serait satisfait par d'autres moyens. Inscrire dans la loi, c'est consacrer des priorités. Autre question posée par le projet

Nous réaffirmons aussi notre opposition ferme et définitive à la légalisation de la vidéosurveillance algorithmique par ce projet de loi. La détection, par logiciel, d'événements et de comportements considérés comme suspects portera une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et à la liberté d'aller et venir des participants.

Le texte de la CMP nous propose d'autoriser de façon pérenne l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par ses empreintes génétiques, afin d'améliorer les contrôles antidopage. En consacrant un caractère durable à ce procédé, la commission mixte paritaire n'a pas pris en compte les réserves émises par la Cnil et la Ligue des droits de l'homme qui dénonçaient déjà en première lecture des tests particulièrement des tests particulièrement intrusifs et dérogeant de façon importante aux principes encadrant les analyses génétiques dans le code civil. Je salue tout de même la tout de même la suppression de l'article 8 , qui prévoyait la présence inopportune des agents des autorités organisatrices exerçant des missions relatives à la sûreté des transports parmi les agents autorisés à visionner les images de vidéosurveillance, ainsi que celle de l'article 2 .

raison pour laquelle le groupe CRCE refuse ce texte, qui ne respecte pas le juste équilibre entre sécurité et protection des libertés et droits fondamentaux et qui n'honore pas l'esprit universel et fraternel des jeux Olympiques. J'espère, madame la ministre, que

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, pour la troisième fois, le Parlement examine une loi permettant de préparer les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Pour la troisième fois, un accord a été trouvé entre l'Assemblée nationale, le Sénat et le Gouvernement, preuve de notre attachement au bon déroulement de cet événement. La recherche de cet accord a permis d'aller plus loin que le projet de loi initial.

Des garanties indispensables ont été maintenues sur les conditions de réalisation de ces tests et un bilan sera remis au Parlement au plus tard le 1 juin 2025.

Il s'agissait de la première recommandation du rapport conjoint de notre commission et de la commission des lois sur les événements survenus au Stade de France le 28 mai 2022, à l'occasion de la finale de la Ligue des champions. Je remercie les présidents François-Noël Le dispositif adopté tient compte des spécificités des compétitions. Il entrera en vigueur le 1 juillet 2024 et s'appliquera donc aux jeux Olympiques et Paralympiques, mais également à la saison 2024-2025 de certains championnats. Nous serons attentifs, madame la ministre, aux dispositions d'application renvoyées au pouvoir réglementaire. Enfin, mon troisième point de satisfaction concerne l'article 14 A qui prévoit que la Cour des comptes remettra au Parlement un rapport d'étape sur le bilan des Jeux avant le 1 octobre 2025. Ce rapport est important : nous avons demandé qu'il fasse notamment toute la lumière sur les dépenses cachées qui auront été engagées par l'État et les collectivités territoriales au travers de la mise à disposition de moyens publics. Si nous sommes vigilants sur cet aspect du bilan des Jeux, c'est que nos débats n'ont pas permis de clarifier pleinement les conditions qui permettront de garantir leur sécurité. Nous avons pu mesurer, à l'occasion de la finale Nous avons pu mesurer, à l'occasion de la finale de la Ligue des champions de mai dernier, les insuffisances du dispositif mis en oeuvre et les difficultés du Gouvernement à reconnaître les erreurs commises.

également révélé le 30 mars dernier que les états-majors des armées envisageaient de préparer des plans de mobilisation de leurs forces pour éviter un scénario catastrophe. La mission d'information sur les jeux Olympiques et Paralympiques de la commission de la culture poursuivra donc ses travaux dans les semaines à venir, afin de lever les interrogations qui demeurent sur l'organisation de cet événement et d'informer les Français.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, j'ai déjà dit à cette tribune mon attachement pour le sport, qu'il soit de haut niveau, mais également amateur, scolaire et universitaire.

ne devrait pas être la promotion d'un « sport business » pensé d'abord comme une économie. Nous allons découvrir sur les chaînes du service public de nombreux sports et athlètes peu connus, mais tout aussi méritants que nos stars médiatisées. Les Kylian Mbappé et autres Antoine Griezmann laisseront la place pour que nous célébrions, le temps de quelques semaines, des champions anonymes de pentathlon moderne, de gymnastique rythmique, de cyclisme sur piste ou encore d'escrime. d'escrime. Pour que nous puissions en profiter sereinement, il faut des lois. Notre Parlement en avait adopté une première le 26 mars 2018. Ce second projet de loi devrait donc achever nos travaux. Sans entrer dans le détail de chacun des articles, je souligne que notre assemblée a apporté un certain nombre d'améliorations, notamment en renforçant des dispositifs juridiques. Je pense par exemple à l'article 11, qui étend l'usage des scanners corporels au contrôle de l'accès aux enceintes dans lesquelles sont organisés certains événements sportifs et culturels.

Elles portent principalement sur les dispositions de l'article 7, au sujet duquel je reprends les mots de notre président Jean-Claude Requier, ici présent La peur d'une société sous surveillance automatisée, à la mode orwellienne, est souvent agitée de manière excessive, mais parfois l'épouvantail se justifie. C'est le cas ici. Nous devons donc faire preuve de vigilance quant à l'utilisation de ces dispositifs vidéo auxquels sont associés des traitements algorithmiques. Ces nouvelles techniques n'ont rien d'anodin. Beaucoup ont indiqué que la ligne rouge de la reconnaissance faciale n'avait pas été franchie ; nous devons néanmoins rester vigilants à toute évolution. Notre groupe est fondamentalement attaché aux libertés, ce qui comprend le respect de l'intimité de chacun, y compris dans l'espace public.

Certes, le dispositif proposé n'est qu'une expérimentation, mais chacun sait ici que l'expérience est le chemin vers la normalisation. J'espère que nous n'aurons pas à le regretter.

Nous espérons néanmoins avoir été entendus et qu'il n'y aura pas de difficulté dans la réaffectation des personnels de sécurité, notamment les compagnies de CRS maîtres-nageurs sauveteurs (MNS), temporairement déplacés pendant les Jeux. Malgré ces remarques, le groupe RDSE votera en faveur de ce texte, avec l'espoir que les jeux Olympiques et Paralympiques soient une réussite avant tout sportive et participent à la concorde universelle.

Si une partie de notre hémicycle a beaucoup reproché à ce projet de loi de n'être dédié qu'à la sécurité, nous pensons pour notre part qu'il était nécessaire, dans un contexte de risque d'attentat, mais également après le fiasco du Stade de France, de tirer tous les enseignements pour ne plus jamais reproduire les mêmes erreurs dans l'organisation de grands événements sportifs internationaux. La panique et le chaos qui ont régné avant la finale de la Ligue des champions, qui devait être un jour de fête pour les amateurs de sport, sont une honte pour notre pays. Il est donc inimaginable de reproduire un tel traumatisme l'an prochain pour des Jeux d'été que la France attend depuis cent ans. Nos athlètes se préparent depuis des années afin d'être prêts pour cette compétition. Nous leur devons, vous leur devez, d'organiser au mieux ces Jeux. Notre pays doit être préparé à accueillir une manifestation aussi exceptionnelle par son ampleur, son périmètre et sa durée. Il s'agit, d'une part, d'accompagner la performance des sportifs et, d'autre part, de garantir des conditions d'accueil dignes pour le grand public. Sur le premier volet, le Sénat a renforcé la réglementation en matière de lutte contre le dopage et facilité l'offre de soins pour les athlètes. Sur le second, relatif

de la commission mixte paritaire autorise une expérimentation, tout en offrant des garanties pour éviter les abus. Aucun système d'identification biométrique n'est autorisé, pas plus que les rapprochements ou mises en relation automatisées avec d'autres traitements de données. Le public sera informé au préalable du traitement des données recueillies. Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, sera régulièrement informé des conditions de traitement et en fera part aux maires des communes concernées, ainsi qu'à la Cnil.

cas de récidive. Des inquiétudes persistent malgré tout en matière de sécurité, par exemple sur la sécurisation des sites de compétition. Alors que le secteur fait face à une pénurie de main-d'oeuvre, les sociétés de sécurité pourraient rencontrer des difficultés pour recruter et former les 22 000 agents, notamment les femmes, nécessaires chaque jour pour assurer la sécurité et le contrôle à l'entrée des sites. Ces inquiétudes commencent à s'ancrer profondément et amènent à s'interroger sur un éventuel recours à l'armée. La semaine dernière, le chef d'état-major des armées confirmait justement, devant nos collègues députés, la mise à disposition de 10 000 militaires en renfort, pour assurer la sécurisation des jeux Olympiques et Paralympiques. Vous-même, madame la ministre, avez évoqué récemment la possibilité de recruter hors de France, peut-être dans des pays francophones.

À ces questions que nous nous posons depuis des mois s'ajoutent de nouvelles inquiétudes. Lors de la première lecture au Sénat, je vous alertai déjà sur les angles morts concernant les volontaires de Paris 2024

au sabotage sur les réseaux sociaux, de la part de militants se revendiquant de l'écologie politique ou de la gauche anticapitaliste. Ils s'opposent à la tenue des Jeux et au principe même du bénévolat et veulent être engagés comme bénévoles pour ensuite déserter ou dégrader des biens. C'est en amont qu'il faut identifier et contrer ces risques d'infiltration par des groupes qui se mobilisent dès maintenant pour gâcher un moment très attendu.

Près de 40 000 bénévoles, plus de 4 millions de téléspectateurs, 4 000 athlètes paralympiques et 10 500 athlètes olympiques : ces chiffres donnent le vertige.

Au fil des débats, nous avons étudié l'ensemble des nombreuses dispositions en matière de lutte contre le dopage, de sécurité, d'adaptation aux territoires d'outre-mer, mais aussi en matière sanitaire. Cette version finale du texte permettra d'assurer le bon déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques sur l'ensemble du territoire. Je me réjouis que la commission mixte paritaire ait conservé une grande partie du ait conservé une grande partie du travail du Sénat. Je pense particulièrement aux dispositions visant à améliorer l'accessibilité des équipements et des épreuves. C'est avec émotion que nous admirerons,

En matière de sécurité, l'organisation des jeux Olympiques en France nous oblige à assurer un haut niveau de protection. Cet événement constituera un véritable défi pour nos forces de sécurité qui devront mener à bien cette mission, en parallèle de celles qui les mobilisent au quotidien. Nous aurons besoin du concours de tous les acteurs. Les agents de sécurité des transports publics seront aussi associés au dispositif. La sécurité privée apportera une aide précieuse, qu'il faudra néanmoins articuler, organiser et contrôler. En plus de cet appui humain, nos services de sécurité pourront compter sur les technologies les plus abouties. Le projet de loi prévoit ainsi l'expérimentation, sur la durée et pour les besoins des Jeux, du traitement algorithmique de la vidéoprotection.

les libertés. Nous sommes fiers d'accueillir cet événement mondial. Nous devons nous donner les moyens d'en faire un vrai moment d'union nationale pour notre pays, qui en a bien besoin en ce moment. Les territoires doivent être pleinement associés à cette aventure olympique.

permettez-moi de profiter de cette prise de parole pour saluer votre action et votre courage politique pour réformer les fédérations sportives- certaines en ont grand besoin. L'éthique du sport doit aussi se retrouver à tous les échelons de la gouvernance sportive. sportive. Nos athlètes olympiques et paralympiques peuvent compter sur notre soutien et nos encouragements. Leur plus grande victoire sera de fédérer l'ensemble des Français

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, « les semaines et les mois passent et l'envolée sécuritaire de ce gouvernement ne retombe pas

Quel est le coeur de ce projet de loi ? Une mise en concordance du droit de la santé pour les questions de dopage ? Une réécriture du code de l'urbanisme en faveur du développement du sport dans nos territoires, dès les Jeux ? Il n'en est rien. Trop peu d'attention a été portée au soutien des fédérations, au sport amateur ou à l'accélération de la pratique sportive pour tous sur l'ensemble de nos territoires. Trop peu d'attention a été portée à l'équilibre des mesures spécifiques et temporaires liées à l'accueil des

C'est l'un de ses aspects les plus remarquables : la mise en oeuvre, sur le temps long, de mesures censées n'être nécessaires qu'au bon déroulement des Jeux. Cette loi va au-delà de l'organisation des JO de Paris. Notre groupe regrette une nouvelle fois une vision sécuritaire débridée et si éloignée des valeurs de l'olympisme. La disproportion des mesures de sécurité- l'un des enjeux de ce texte -cache de réelles atteintes aux droits des personnes, qui s'inscrivent bien au-delà du temps des Jeux. Comme j'ai pu le dire, tout ce déploiement de la vision sécuritaire et le recours massif et presque indifférencié à la vidéosurveillance augmentée

Dans une période où le droit de manifester subit certaines attaques, au moment où le ministre de l'intérieur s'en prend à la Ligue des droits de l'homme, à l'heure où le porte-parole du Gouvernement affirme « qu'il peut y avoir des arrestations faites pour contrôler », notre vigilance sur de tels outils doit être maximale. C'est bien une vision sécuritaire et technologique qui se dévoile et que nous jugeons d'autant plus néfaste et inefficace qu'elle obère complètement la réalité du terrain, où le recrutement la formation des agents de sécurité n'ont pas été anticipés. Nous allons manquer de personnel public et privé. La Cour des comptes estime qu'il faudrait employer entre 22 000 et 33 000 agents de sécurité privée par jour pour véritablement sécuriser l'ensemble des épreuves. Ces chiffres dépassent largement les capacités disponibles dans les entreprises de la région et du pays. La crainte de voir sur le terrain des gens peu formés intervenir dans le cadre d'événements d'une telle ampleur fait ressurgir le spectre du fiasco du Stade de France.

les déclarations et actions du Gouvernement démontrent le déni dans lequel il s'enferme, manquant l'occasion de faire progresser les techniques du maintien de l'ordre et de la gestion des flux de population. Les modifications apportées quant au recrutement dérogatoire des étrangers titulaires de permis de séjour ou de titres étudiants montrent le manque d'anticipation et la précipitation dans laquelle l'organisation de la sécurité d'un tel événement se fait. peut nourrir sur la mise en place de mesures de sécurité disproportionnées, rien dans le texte ne vient éloigner l'hypothèse d'une explosion des coûts comparable à celle de l'expérience londonienne.

L'ambition de ce texte est simple, mais elle est de taille : faire de ces Jeux un succès populaire en relevant le défi de leur organisation et en assurant la sécurité- y compris sanitaire -des athlètes, des bénévoles et des spectateurs venus du monde entier.

L'article 7 de ce projet de loi, qui prévoit l'expérimentation de la vidéosurveillance augmentée par l'intelligence artificielle, en est certainement l'exemple le plus frappant. Le dispositif que nous nous apprêtons à voter est, me semble-t-il, de nature à rassurer celles et ceux qui, comme nous, sont profondément attachés au respect des droits fondamentaux et des libertés publiques.

Nous nous réjouissons que la commission mixte paritaire ait préservé les apports du Sénat, plus particulièrement les garanties entourant la phase de développement des traitements algorithmiques.

Nous notons par ailleurs avec satisfaction que le texte prévoit un meilleur encadrement des données d'apprentissage, qui ne pourront être utilisées que pendant une durée maximale de douze mois à compter de l'enregistrement des images. qui concerne la sécurité des manifestations sportives, le groupe RDPI accueille favorablement la suppression de la disposition tendant à délictualiser les infractions prévues à l'article 12 lorsque les faits n'ont pas été commis en réunion ou en récidive. Cette disposition, introduite par le Sénat, était à nos yeux disproportionnée. Il apparaît plus raisonnable de sanctionner les primo-délinquants isolés par une amende contraventionnelle de Je tiens à remercier nos collègues députés d'avoir introduit des dispositions nouvelles, qui contribueront à la bonne organisation des jeux Olympiques et Paralympiques. Je pense notamment à la possibilité donnée aux vétérinaires d'exercer la médecine et la chirurgie dans le cadre de la préparation et du déroulement des épreuves équestres. Je pense également à la clarification du régime applicable aux contrôles antidopage de nuit. La facilitation de l'embauche des étudiants étrangers comme agents de sécurité privée va dans le bon sens, de même que l'encadrement du régime des interdictions administratives de stade. Permettez-moi, en outre, de me réjouir que les dispositions relatives aux outre-mer soient inscrites en dur dans le texte. Parmi les rares points de désaccord entre nos deux chambres figuraient les dispositions relatives à l'application des règles antidopage en Polynésie française. À cet égard, le groupe RDPI se félicite du rétablissement de la disposition prévoyant l'homologation des peines de prison prévues par les deux lois du pays du 26 novembre 2015. La suppression de cette disposition aurait en effet créé un vide juridique incompatible avec l'objectif visé, à savoir le renforcement de l'efficacité de la lutte contre le dopage en vue des épreuves olympiques de surf. Le groupe RDPI votera donc avec enthousiasme en faveur de ce texte, qui contribuera à faire des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 un succès sportif et une grande réussite française. Nous vous proposons en conséquence d'emboîter le pas à l'Assemblée nationale qui a adopté, hier, ce projet de loi.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes à 471 jours du début des jeux Olympiques et c'est la fin de la préparation législative de cette échéance. Le projet de loi de mars 2018 avait été adopté à l'unanimité, témoignant ainsi de la bonne volonté de l'ensemble de ceux qui siègent sur ces travées dans l'optique de la réussite de Paris 2024. Ce projet de loi aura été moins consensuel, tant dans cet hémicycle qu'à l'Assemblée nationale. Avec mes collègues du groupe socialiste- je pense notamment à Jean-Jacques Lozach, Corinne Féret ou Sylvie Robert -, nous avons fait de notre mieux pour apporter notre pierre à l'édifice. En effet, nous souhaitons tous ardemment la réussite de ces Jeux,

parce qu'ils représentent pour la jeunesse française une chance rare d'accueillir le monde. Bon nombre de mesures très utiles sont présentes dans les vingt-quatre articles de ce projet de loi. Ainsi, les adaptations nécessaires en matière d'offre de soins et de formation aux premiers secours sont compréhensibles. On perçoit bien la nécessité d'avoir un centre de santé au sein du village olympique, tout comme la possibilité de former davantage de monde aux premiers secours. En première lecture, nous nous étions félicités du contenu de ce texte concernant la lutte contre le dopage. Nous avions accepté plusieurs mesures relatives à la mise en conformité du régime de la vidéoprotection avec le droit européen sur la protection des données. Mais le fameux article 7, relatif à la vidéosurveillance algorithmique, et la tonalité générale du texte, très sécuritaire, nous avaient refroidis. Les débats en commission mixte paritaire ont été francs et je tiens à saluer le travail de notre collègue rapporteur Mme Canayer. La commission mixte paritaire a permis plusieurs avancées notables avancées notables : suppression de l'article 8 , qui tendait à ouvrir un peu trop grandes les portes du centre de commandement opérationnel de la préfecture de police ; suppression de l'article 12 , qui prévoyait l'aggravation des sanctions pénales applicables aux auteurs de violences commises dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive ; enfin, limitation

de l'article 1 relatif à la campagne des violences sexistes et sexuelles sur les sites du village des athlètes et du village des médias. Nous ne voyons pas en quoi cet article posait problème. Il aurait été avantageux de le maintenir. Nous regrettons aussi l'augmentation à douze mois de la durée de conservation des images comme données d'entraînement des algorithmes. Il ne nous Il ne nous semblait pas illogique de s'aligner sur le droit commun sur ce point. Si le Conseil constitutionnel valide ce dispositif, ce qui reste à vérifier, j'espère que les organisateurs de la Coupe du monde de rugby préviendront les spectateurs que leurs images serviront à entraîner les algorithmes pour La suppression de la référence au 19.6 de SecNumCloud a été justifiée par le fait qu'aucune entreprise française ne détenait ce label. Toutefois, la partie de l'article 7 issue de cet amendement ne concernait que la protection vis-à-vis du droit extraterritorial. J'aimerais revenir sur les sujets qui n'ont pas pu être abordés par voie d'amendement, mais qui occupent et occuperont le débat public la privatisation du réseau de bus, la taxe de séjour dans les hôtels de luxe des villes hôtes, le travail le dimanche dans les communes concernées par les Jeux ou l'affectation de renforts humains pour assurer la sécurité des jeux Olympiques, qui a déjà été évoquée par plusieurs de nos collègues- Jean-Pierre Sueur, auteur d'une proposition de résolution sur l'article 45 de la Constitution, Nous étions entrés dans la discussion parlementaire de manière constructive, en souhaitant, j'y insiste, la réussite des Jeux. Le texte déposé par le Gouvernement n'était pas parfait, la discussion en commission et dans l'hémicycle n'a pas levé tous nos doutes. Des inquiétudes légitimes autour de l'article 7 ont beaucoup crispé. Il est d'ailleurs curieux de constater que l'intelligence artificielle,

Notre vote d'abstention s'explique par cet article 7. Même si les Jeux doivent être une réussite et que ce texte y contribue, le pas franchi à la faveur de la mise en oeuvre de cette vidéosurveillance intelligente est inopportun, voire dangereux.